Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, toutes les minutes, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique est déversé dans les mers et les océans, bien triste réalité

Cette proposition de loi présente des mesures préventives et ciblées qui permettraient, dès à présent, de diminuer cette contamination diffuse, invasive et persistante. Je tiens à remercier la rapporteure, ma collègue Martine Filleul, de son implication et de son travail, qui ont permis d'enrichir ce texte.

Le plastique est devenu l'un des maux de notre siècle, une véritable bombe à retardement. La polyvalence des plastiques les a rendus omniprésents dans notre quotidien. Paradoxalement, alors qu'ils avaient été conçus pour être résistants, ils sont devenus le produit star de l'usage unique et du tout jetable. La production de matière plastique connaissant aujourd'hui une croissance exponentielle, les usages se sont multipliés ces dernières années. Au rythme actuel, si l'on ne fait rien, cette production devrait doubler d'ici à 2050. S'ajoute à cela le fait qu'on estime aujourd'hui que 81 % des plastiques mis en circulation deviennent des déchets en moins d'une année d'utilisation. Il y a une multitude de plastiques. Chacun d'entre eux a sa formulation, qui consiste en un polymère de base- polyéthylène, polypropylène, polystyrène, par exemple -auquel on a ajouté des charges- du mica, ou encore des plastifiants, comme les phtalates, et des additifs tels que colorants, anti-UV, antioxydants ou retardateurs de flamme. L'appellation générique de « plastique » est en cela l'arbre qui cache la forêt des centaines de formulations possibles et différentes. Chaque industriel met au point une formulation qui convient à l'usage, à l'apparence et aux propriétés spécifiques de l'objet qu'il souhaite fabriquer. L'élément central et qui explique son usage exponentiel est le triptyque faible coût, légèreté, résistance. Le plastique ne fait pas exception à la règle : il a les défauts de ses qualités. Comme il est peu coûteux, on le veut vierge plutôt que recyclé ; comme il est léger, il s'éparpille dans la nature ; comme il est résistant, il va y persister des il va y persister des centaines d'années, car le plastique ne se décompose pas, mais va seulement se fragmenter. C'est à ce constat que nous nous heurtons. Ce que nous découvrons jour après jour, c'est combien cette pollution par le plastique est diffuse et insidieuse. Elle ne se limite pas aux déchets visibles que sont les macroplastiques, mais consiste aussi en microplastiques et même en nanoplastiques. Les microplastiques proviennent soit de la fragmentation des plastiques, soit d'un ajout intentionnel, comme celui de microbilles dans les cosmétiques, les peintures, ou encore les détergents, ce que les consommateurs ignorent d'ailleurs Pour finir de dresser l'état des lieux, je veux évoquer les images marquantes et choquantes d'animaux étouffés par ingestion, ou enchevêtrés dans du plastique. Oui, la biodiversité se meurt de notre inaction. On dénombre plus d'un million d'oiseaux et 135 000 mammifères tués tous les ans par le plastique. Non moins choquante, l'extrême pollution de la Méditerranée lui vaut de se hisser au triste rang de mer la plus polluée au monde. Elle ne reçoit pas moins de 600 000 tonnes de déchets de plastique par an. À vrai dire, nos mers sont devenues des déversoirs. Il existe cinq gyres de plastique dans les océans. On parle même de « continent plastique », véritable soupe de microplastiques. Plus récemment, des recherches ont relevé la présence de microfibres dans les glaces de l'Everest, des microplastiques dans les eaux de l'Antarctique et même dans l'air au sommet du pic du Midi. quelques chiffres éloquents : 200 millions de tonnes de déchets de plastique se sont accumulées dans les océans à ce jour, 8 millions étant déversés chaque année. En France, 80 000 tonnes sont rejetées chaque année sur le littoral et dans la nature.

Si les microplastiques ingérés sont souvent excrétés, il n'en est pas de même pour les nanoplastiques, qui pourraient franchir par translocation les barrières cellulaires, ce qui est pour le moins inquiétant. Dans le cas où le déchet n'est pas excrété, par exemple un bouchon de plastique dans l'estomac d'un oiseau, il va y séjourner, créer de la satiété, affaiblir l'animal et finir par le tuer. Ces perspectives de contamination de l'ensemble de la chaîne alimentaire et du vivant sont déjà alarmantes, alors même que tous les effets n'ont pas encore été mesurés. Dans l'environnement le plastique va connaître trois types d'échanges. Premièrement, il se charge des polluants hydrophobes, comme les polychlorobiphényles (PCB) et les hydrocarbures, qu'il rencontre lors de son séjour dans l'eau, l'air ou les sols. Ainsi, en cas d'ingestion, un animal va absorber non seulement le plastique, mais aussi les polluants dont il s'est chargé.

Par exemple, des années après le tsunami de Fukushima de 2011, des espèces invasives transportées par des plastiques japonais ont été répertoriées aux États-Unis. Cette colonisation biologique donne par ailleurs au plastique une odeur qui leurre les animaux, ces derniers le confondant avec de la nourriture. Enfin, troisième type d'échange, les plastiques de nouveau les plastifiants et les additifs dès que leur surface s'abîme en se fissurant, ou lorsqu'ils se fragmentent. Certains de ces composés sont aussi des perturbateurs endocriniens, qui affectent durablement, même à très faibles doses, le système nerveux, la fertilité ou encore le développement cérébral des espèces vivantes. Vous comprendrez sans peine que ces matières plastiques nuisent de façon irréversible aux écosystèmes marins et terrestres, portant ainsi atteinte à la biodiversité. la mise en place de politiques publiques de sensibilisation, de prévention et, récemment, d'interdiction ne suffit pas à endiguer le flux et, surtout, l'accumulation de déchets dans l'environnement.

comme il est nécessaire de sensibiliser le consommateur à la portée de ses actes. Cette proposition de loi répond donc à une urgence qui nous impose d'agir concrètement et de commencer à endiguer ces arrivées de plastique dans l'environnement. Préserver notre environnement et notre santé est l'affaire de tous implique non seulement une prise de conscience collective, mais aussi des politiques publiques volontaristes et des mesures législatives fortes. La parole

Je me réjouis d'avoir retrouvé sur cette proposition de loi le même état esprit volontariste et constructif. Je remercie notamment pour leur sens du dialogue la rapporteure de la loi AGEC, Mme Marta de Cidrac, et le président de la commission, M. Jean-François Longeot.

tendant à changer l'intitulé de la proposition de loi de manière à mieux l'articuler avec son objet : la lutte contre la pollution plastique, plutôt que la lutte contre le plastique. Ce texte vise bien à s'attaquer à la pollution induite par ce matériau, plutôt qu'à cette matière elle-même. Cette précision faite, j'évoquerai les articles de la proposition de loi initiale, ainsi que les amendements sur ces articles qui ont été adoptés en commission. L'article 1 vise à renforcer le cadre juridique relatif aux fuites de granulés de plastique dans l'environnement, introduit dans l'article 83 de loi AGEC sur l'initiative du Sénat. Les rejets annuels dans l'environnement de ces granulés sont estimés, à l'échelle européenne, à 25 000 tonnes. Il est donc urgent de prévenir la fuite de ces granulés qui s'accumulent sur nos littoraux, dans nos mers et dans nos océans. océans. Afin de s'adapter à la rédaction de l'article 83 de la loi AGEC et de tenir compte du projet de décret d'application, la commission a adopté un amendement de réécriture de l'article 1 à contraindre les sites concernés à déclarer annuellement les pertes et fuites de granulés et à mettre en place des systèmes d'information par voie d'affichage afin de les prévenir. L'article 2 vise à interdire l'ajout intentionnel de microbilles de plastique dans les détergents. Je rappelle que les rejets annuels de ces plastiques s'élèvent à 36 000 tonnes à l'échelle européenne. Afin de laisser un délai raisonnable aux producteurs pour retirer les produits mis sur le marché et modifier leurs procédés de fabrication à grande échelle, un amendement a été adopté visant à prévoir une entrée en vigueur légèrement différée au 1 juillet 2022.

Pour autant, la commission a estimé nécessaire de clarifier le droit en vigueur ; elle a donc adopté cet article. Enfin, l'article 4 prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux de l'utilisation dans l'industrie textile de fibres de plastique pouvant être à l'origine de microfibres dans l'environnement. J'en viens maintenant aux éléments de débat additionnels qui ont nourri nos travaux en commission. La commission a tout d'abord introduit un article encadrant l'usage des granulés de plastique utilisés sur les terrains de sport synthétiques. Ces granulés se dispersent dans la nature à raison de 50

Deux solutions sont proposées dans un rapport de l'Agence européenne des produits chimiques (AEPC) qui devrait paraître très prochainement : une interdiction ou la mise en place de mesures techniques de confinement au niveau des terrains de sport. Ces solutions seront prochainement soumises à l'arbitrage de la Commission européenne et des États membres. Les mesures de confinement proposées n'offrent qu'une garantie limitée en matière environnementale, en comparaison avec une restriction d'usage. De surcroît, rien n'indique que ces mesures de confinement seront moins coûteuses à mettre en place pour les collectivités territoriales. Enfin, des alternatives aux granulés de plastique pourraient être développées à l'échéance visée, sous la forme de liège ou de noyaux d'olives broyés. C'est pourquoi la commission a adopté un amendement visant à ce que l'emploi de ces granulés soit interdit pour les nouveaux terrains de sport mis en service à compter du 1 mars 2026. Nous invitons le Gouvernement à retenir cette position dans le cadre des négociations qui se dérouleront dans les mois à venir au niveau européen. Cette position est suffisamment pragmatique pour donner une perspective aux collectivités territoriales, car elle s'appliquera uniquement aux nouveaux terrains de sport.

Producteur de 600 millions d'emballages à usage unique par an, le marché de la restauration livrée connaît une forte croissance- +30 % -, accélérée encore par la pandémie de covid-19. Le Gouvernement, pour répondre à ce problème, a annoncé en février 2021 la signature d'une charte pour les acteurs du secteur, afin de réduire les déchets d'emballages.

Ce sujet pourra faire l'objet d'approfondissements dans le cadre des travaux que nous mènerons sur le projet de loi Climat et résilience.

la pollution plastique est un fléau pour la nature, les écosystèmes et la santé humaine. C'est un fléau de notre époque, de notre temps : en un siècle à peine, le plastique est devenu aussi courant que le ciment et l'acier

comme ailleurs, le temps des discours est révolu : il nous faut maintenant agir concrètement et avec volontarisme, dans la vie quotidienne, dans les usines, les supermarchés et les restaurants, jusque dans les

le compte de l'Opecst, démontre que l'ensemble de la représentation nationale a intégré cette urgence à agir sur le plastique. Je tiens également à saluer le travail de Mme la rapporteure,

Votre texte démontre aussi que la lutte contre les plastiques est une responsabilité collective qui engage chacun d'entre nous, jusque dans nos habitudes quotidiennes.

polyvalents et pratiques, les plastiques connaissent un essor continu depuis les années 1950. En France, près de 5 millions de tonnes sont produites par an, soit 70 kilogrammes par habitant.

On retrouve des microplastiques jusque dans notre alimentation : chacun d'entre nous consommerait ainsi l'équivalent de cinq grammes de plastique par semaine. Certains de ces matériaux contiennent des additifs dangereux, tels que des perturbateurs endocriniens, et nous savons peu de chose sur les effets à long terme sur l'organisme de l'ingestion régulière de microplastiques. Plusieurs

Elle prévoit l'encadrement des pertes et des fuites de granulés de plastique industriels, l'interdiction de l'ajout intentionnel de microbilles dans les détergents et de l'emploi de granulés de plastique sur les terrains de sport synthétiques, responsables à eux seuls, en Europe, d'un rejet annuel de 16 000 tonnes de plastique. L'article L'article 3 punit les lâchers intentionnels de ballons de baudruche en plastique, si ces derniers retombent dans un lieu dont le propriétaire n'a pas donné son accord. La commission a satisfait l'amendement que j'avais déposé en revenant à la version antérieure du texte, supprimant ainsi le renvoi explicite à un régime de sanction, que j'estimais excessif et potentiellement inapplicable.

qui se dispersent notamment les eaux usées. C'est une question pour laquelle une réflexion serait bienvenue. Ce texte offre des avancées certes utiles, mais limitées. Il faut aller plus loin et systématiser la lutte contre cette forme de pollution. Le rapport de notre collègue Martine Filleul donne l'exemple du secteur de la livraison de repas : il connaît un véritable boom, accentué par la pandémie de covid-19, et représente à ce jour plusieurs centaines de millions de repas par an. Le Gouvernement a annoncé, en février dernier, la signature d'une charte par les acteurs du secteur afin de réduire les déchets d'emballages. Celle-ci devrait être contraignante, et insister sur le réemploi des contenants, qui, selon des études, n'est pas plus coûteux que l'utilisation d'emballages jetables. De même, une occasion a été manquée avec les déchets liés à la pandémie de covid-19 : masques, visières de protection et gants, trop souvent, ne font pas l'objet de tri et sont incinérés ou abandonnés sur la voie publique ou dans la nature. Pourquoi ne pas mettre en oeuvre les alternatives durables existantes ? Certaines entreprises désinfectent ces plastiques par ultraviolets puis les transforment en granulés pour fabriquer de nouveaux objets, ou les broient en flocons et les mélangent à une résine afin d'obtenir un matériau lui-même recyclable. Les discussions autour du projet de loi Climat et résilience nous permettront de poursuivre la réflexion. Pour l'heure, le groupe du RDSE votera dans sa grande majorité cette proposition de loi, qui apporte sa pierre à l'édifice de la lutte contre la pollution plastique. La parole

stratégie adoptée, celle des « petits pas ». Nous déplorons ainsi des mesures certes utiles, mais qui, sans changement de paradigme, ne réduiront qu'à la marge le problème, sans en traiter les racines. En effet, il est vain d'imaginer promouvoir réellement l'économie circulaire et la limitation des déchets de plastique, sans agir de manière plus forte sur notre modèle de production, en appréhendant ces questions uniquement sous l'angle de la réglementation de la consommation, de la production des déchets et de leur traçabilité. Nous pensons, bien au contraire, qu'il faut en finir avec l'ordre cannibale qui pille et exploite ! Il convient ainsi de repenser l'ensemble de la chaîne de production. Qui décide Comment produit-on et pour qui ? Sous quel contrôle démocratique et citoyen ? Ces questions sont trop sérieuses pour être laissées à la main des lobbies ou des accords de libre-échange- vaste sujet

pour partie, un amendement déjà déposé par la sénatrice Préville lors de l'examen de la loi AGEC. Nous le soutiendrons une nouvelle fois ! Le rapport demandé à l'article 4 nous paraît particulièrement opportun, considérant que la pollution par le liée aux textiles constitue une source majeure de dégât environnemental. La fondation Ellen MacArthur décrivait en 2015 une fuite de 500 000 tonnes par an de ces fibres minuscules, sur une production totale de 53 millions de tonnes de textiles. Il convient donc d'avancer sur ces questions.

alternatives naturelles à la production de textile à base de plastique. Ce problème repose la question de la maîtrise des enjeux de production et de limitation de la consommation. En outre, nous sommes en accord avec l'article inséré lors de l'examen en commission portant interdiction des granulés pour les terrains de sport.

pour limiter le plastique à usage unique, que le Gouvernement a malheureusement fait le choix d'écarter, réduisant encore un peu plus la portée d'un texte pourtant attendu.

nous avons profité des bienfaits des hydrocarbures jusqu'à la lie. L'exploitation du pétrole s'est accompagnée de progrès considérables : n'oublions pas qu'elle a permis une élévation sans précédent du niveau de vie au cours du XX siècle Il en va de même des produits dérivés du pétrole, au premier rang desquels figure le plastique. Le plastique a été une formidable invention, il a changé nos vies, au point de devenir le matériau miracle de presque toutes les industries. Mais nous en avons abusé. Notre rapporteure, dont je salue l'excellent travail, l'a rappelé : le plastique menace aujourd'hui la santé humaine et l'ensemble de l'écosystème planétaire. Face à ce constat, nous ne pouvons que revoir nos choix technologiques et économiques. Face au plastique, il n'y a qu'une seule solution durable : réduire radicalement sa production ! Blâmer l'incivilité de l'utilisateur et prôner le recyclage revient en réalité à se défausser. Certes, si du plastique se retrouve dans la nature, c'est parce qu'on l'y jette. Mais c'est surtout parce que l'industrie en déverse chaque année des milliards de tonnes sur le marché. Le recyclage engendre mécaniquement la production de nouveaux plastiques.

La pollution due aux ballons de baudruche, couverte par l'article 3, est sans doute plus anecdotique ... Je salue l'amélioration apportée au texte par la commission, qui a introduit un article interdisant les granulés de plastique dans la fabrication des terrains de sport synthétiques. Bien sûr, tout cela n'est pas neutre économiquement. Le plastique représente beaucoup d'emplois sur nos territoires. Mais ces emplois peuvent être sauvés parce que le secteur peut effectuer sa transition De la même manière que les pétromonarchies et Total ont massivement investi dans les nouvelles énergies, nombre d'industriels du plastique investissent déjà dans de nouveaux matériaux. La bonne nouvelle, c'est que le secteur a les moyens d'investir dans sa transition. Aidons-le à faire sa mue en allant demain encore plus loin dans la lutte contre le plastique à usage unique et le suremballage ! En attendant, l'immense majorité du groupe UC votera en faveur de la présente proposition de loi.

chers collègues, permettez-moi de remercier notre collègue Angèle Préville d'engager de nouveau le débat sur la question de la pollution par le plastique, à la suite de son rapport pour le compte de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Déjà, à cette époque, les débats avaient été nourris et constructifs, et nous avions su enrichir le texte du Gouvernement : 164 amendements avaient ainsi été adoptés en commission et 222 en séance publique. Le travail parlementaire avait plus que jamais fait ses preuves à cette occasion. J'étais rapporteure de ce texte pour le Sénat et c'est pour moi, encore aujourd'hui, un sujet de fierté ! Plusieurs des dispositions concernaient la lutte contre la pollution par le plastique. Mme la ministre de la transition écologique a d'ailleurs annoncé avoir signé le décret sur la réduction des emballages en plastique à usage unique d'ici à 2025- c'est une excellente nouvelle

le temps qui m'est imparti, je ne pourrai m'arrêter que sur quelques articles. L'article 1, tout d'abord, est relatif à l'encadrement des pertes et des fuites de granulés de plastique industriels. La loi AGEC, en son article 83, prévoit déjà des avancées sur ce point- cette disposition était d'ailleurs l'oeuvre d'un amendement de Mme Préville. La consultation publique portant sur le décret d'application de cet article s'étant achevée au début du mois, la publication ne saurait se faire attendre.

2, quant à lui, vise à interdire l'ajout intentionnel de microbilles dans certains biens. Là encore, le sujet a déjà été débattu dans cet hémicycle. Le Sénat avait d'ailleurs pris des dispositions permettant de faire financer par les producteurs des opérations de traitement de la pollution des eaux.

question d'affaiblir une filière française qui représente 200 000 emplois, ce qui nous obligerait à importer du plastique ; c'est une dimension essentielle à prendre en compte. Toutefois, n'oublions pas que la loi n'est pas le seul instrument de lutte contre la pollution par le plastique ! Nous avons tous pu le constater, depuis mars 2020 et le début de la crise pandémique, le plastique a pris une place importante dans nos vies les masques et autres équipements de protection nécessaires, ainsi que les emballages se sont multipliés. Que faire face à ce phénomène ? Au-delà du volet législatif, deux leviers peuvent être activés. Le premier est relatif à la prévention auprès des consommateurs et à l'évolution des habitudes. Le second concerne la recherche et le développement de matériaux substituables au plastique. Cette recherche évolue dans de très nombreuses directions ; c'est elle qui permettra une transition et une adaptation de notre société face à la pollution par le Tout est question d'équilibre : il faudra toujours veiller à ce que ces alternatives ne soient pas plus mauvaises, mais aussi à accompagner les filières dans cette transformation à court, moyen et long terme, au-delà du plan de relance qui court jusqu'en 2022. Aussi, appuyons-nous sur les initiatives existantes pour réduire la pollution par le plastique, et prenons en considération la dynamique européenne, essentielle sur ces questions

la lutte contre la pollution par le plastique sera l'un des grands enjeux de notre siècle. Ce matériau a pourtant grandement facilité notre vie et reste parfois incontournable, particulièrement pour les dispositifs médicaux comme les poches de sang.

propres doivent être poursuivies. Aussi, j'accueille très positivement l'interdiction à l'horizon de 2026 de l'utilisation de granulés de plastique dans les installations de terrains de sport synthétiques. Grâce aux solutions de remplacement, elle aura un effet significatif. Je salue également l'interdiction de microbilles de plastique dans les détergents. C'est d'autant plus important qu'elles sont très souvent directement évacuées dans nos canalisations, avec les conséquences que l'on connaît

créer un cercle vertueux autour d'un plastique moins polluant et utilisé seulement dans les cas nécessaires. Cela semble cohérent avec la réalité actuelle et les enjeux environnementaux.

C'est pourquoi je considère comme cruciale la discussion ouverte en commission par notre rapporteure sur les contenants réutilisables et consignés dans le domaine de la livraison de repas. Là encore, les industriels se montrent ouverts, comme c'est souvent le cas. Ils sont conscients des enjeux et des transformations à venir. Notre rôle, en tant que législateurs, est de les accompagner et de les encadrer dans cette transition nécessaire.

La qualité de l'eau est excellente dans beaucoup de nos départements- ressortons les carafes en verre ! Nos océans, nos mers, nos forêts, nos villes et notre biodiversité meurent de la pollution des bouteilles en plastique

sont effectivement recyclés ... Les priorités politiques devraient donc viser à réduire la consommation et encourager des modèles commerciaux fondés sur le réemploi et développer le recyclage. Le coût de la pollution par le plastique n'étant pas supporté par les acteurs qui tirent profit de sa production ou de son utilisation, il est moins coûteux de rejeter les déchets dans la nature que de gérer leur fin de vie ! Cette absence de responsabilité a conduit à une production insoutenable et à une pollution croissante- le rapport parle de « bombe à retardement » -, avec le danger des microplastiques et des nanoplastiques invisibles et encore mal connus. Nous devons réguler et maîtriser ce grand déversoir

avec des conséquences dramatiques pour la biodiversité. Se fondant sur ce constat alarmant qui dépasse largement nos frontières, l'Union européenne n'est pas restée inactive. Elle a ainsi diligenté l'Agence européenne des produits chimiques qui, depuis 2019, a proposé une restriction de grande ampleur relative aux microplastiques présents dans les produits mis sur le marché dans l'Union européenne. La proposition de loi présentée par Mme Préville s'inscrit dans cette volonté de réduction. Elle fait suite au projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

respectivement autrice et rapporteur d'une proposition de loi du groupe RDPI : ils ont alerté dès 2018 sur les conséquences sanitaires et environnementales de l'utilisation

de l'examen du projet de loi Climat et résilience, et je l'espère, avec le même esprit collectif. Enfin, au-delà de notre rôle de législateur, l'Europe agit également. Réjouissons-nous que la France,

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, il y a un peu plus d'un an, nous votions ici même, au Sénat, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, la loi AGEC. Le groupe socialiste et le Sénat dans son ensemble avaient su rehausser les ambitions de ce texte. Au nom de mon groupe, j'avais défendu un amendement conservé dans la rédaction finale de la loi tendant à introduire un principe général selon lequel toutes les politiques publiques doivent fixer des actions à mettre en oeuvre pour lutter contre la pollution causée par les plastiques dans l'environnement et réduire l'exposition des populations aux particules de plastique. plastique. En tant que premier producteur européen de déchets de plastique, la France doit en effet avoir une véritable ambition en matière de lutte contre cette pollution. Sans infléchissement de nos modèles économiques, cette production devrait doubler d'ici à 2050. La présente proposition de loi, présentée par notre collègue Angèle Préville, dont on connaît la ténacité sur ce sujet, s'inscrit dans cette logique en apportant de précieuses avancées juridiques et en ouvrant une nouvelle séquence au Sénat, en amont de l'examen du projet de loi Climat et résilience. Son récent rapport réalisé au nom de l'Opecst est extrêmement convaincant quant à l'urgence d'une action contre cette pollution pollution massive, qui conduit aujourd'hui les scientifiques à rebaptiser l'anthropocène « plasticocène ». Fondé sur ce constat aussi troublant qu'accablant, le présent texte contient des mesures concrètes et ciblées qui ont déjà été largement présentées. L'article 1 vise ainsi à encadrer les pertes et fuites de granulés de plastique industriels, les célèbres « larmes de sirènes » que l'on retrouve quotidiennement sur nos plages jusque sur les bords de la Loire- que je connais bien -et même sur les bords du Der. La disposition proposée est très utile, car elle couvre certains angles morts qui persistent dans le décret en préparation. Dans la même veine, l'interdiction de l'introduction intentionnelle de microbilles de plastique dans les détergents prévue à l'article 2 est de bon sens. Nous avions d'ailleurs voté cette disposition ici même, mes chers collègues, lors de la première lecture du projet loi AGEC. Enfin, l'article 4 met en exergue une problématique aiguë qui demeure un impensé industriel : les microfibres de plastique contenues dans les textiles. Cette demande de rapport est un pavé dans la mare pour une industrie qui a longtemps fermé les yeux sur son impact environnemental. Le rapport de l'ONG Changing Markets Foundation publié le 2 février dernier démontre que l'utilisation du polyester dans les vêtements à bas coût a doublé en vingt ans. Le relargage des fibres textiles dans l'environnement est ainsi évalué à l'échelon européen entre 18 000 et 46 000 tonnes par an. Ce que l'on nomme la, ou « mode jetable », doit sérieusement prendre en compte cet état de fait. je tiens à remercier notre rapporteure Martine Filleul de la qualité de son rapport et de ses propositions qui ont encore permis d'améliorer ce texte. L'unanimité avec laquelle notre commission a voté celui-ci est de bon augure et démontre que, sur ces questions, le Sénat est capable de dépasser les clivages partisans pour l'intérêt général. J'espère que le Gouvernement, par votre voix, madame la secrétaire d'État, se ralliera à ces dispositions très étayées et vitales pour « déplastiquer » progressivement, mais sûrement, notre économie, et surtout notre environnement. La parole

Les industriels ont répondu présent en fournissant surblouses, visières et autres matériels essentiels en temps de crise sanitaire. Ce secteur d'activité s'efforce également de répondre aux ambitions environnementales et écologiques, en favorisant les meilleures solutions d'emballage éco-efficaces et performantes, en rationalisant l'usage du plastique et en évoluant vers la mise en place de filières de valorisation des déchets. Les professionnels de la filière plasturgie intègrent aujourd'hui les technologies et les compétences de l'économie circulaire. Par exemple, en Haute-Loire, le groupe Coveris flexibles France, qui détient l'un des plus gros sites de production industrielle du secteur de la plasturgie de mon département, a investi 7 millions d'euros pour répondre aux nouvelles attentes du marché et aux contraintes réglementaires. À l'horizon de 2023, le groupe entend proposer 85 % de produits recyclables, issus pour 45 % de nouvelles productions à base de matières plastiques recyclées, de matière monomatériau et de papier.

Seulement 32 % des mesures sont actuellement appliquées de manière effective, la majeure partie des décrets d'application étant encore en cours de rédaction, en raison de l'ampleur des transformations proposées dans ce texte de loi. Au-delà de la mise en oeuvre, il est important de souligner qu'une transition écologique réussie ne peut se faire sans une certaine stabilité du contexte réglementaire. Même si nous approuvons les objectifs de lutte contre la pollution, par le plastique, mais toutes les formes de pollution, nous constatons que la présente proposition de loi ne fait qu'agiter le totem du plastique alors que nous avons besoin d'apaisement pour avancer concrètement sur ce sujet. nous pensons qu'il faut adopter une approche plus pragmatique et liée à l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception des produits pour qu'ils soient recyclables à la collecte de ces mêmes produits en fin de vie pour qu'ils soient recyclés, afin qu'aucun plastique ne se retrouve dans l'environnement. Au lieu de multiplier les interdictions, mes chers collègues, aidons nos industriels à aller plus loin en matière de recherche et de développement pour intégrer les filières dans l'économie circulaire pour produire de façon plus durable, plutôt que de les faire disparaître,

le plastique, ou plutôt les plastiques sont présents dans la quasi-totalité des produits que nous utilisons au quotidien : automobile, sport, jardinage, jouets électroniques, cosmétiques- la liste est longue. Ce matériau a permis d'améliorer la conservation des aliments et la lutte contre le gaspillage alimentaire, de sécuriser le secteur médical, de renforcer l'isolation et l'efficacité énergétique ... Je pourrais décliner à l'infini ses apports bénéfiques. Pourtant, nous sommes réunis cet après-midi pour évoquer la pollution causée par le plastique, qui est aussi une réalité. Les chiffres sont édifiants : selon l'ONU, ce sont, chaque seconde, pas moins de 17 tonnes de plastique qui sont déversées dans nos océans, dont 80 % proviennent de déchets abandonnés sur terre.

La France possède le deuxième espace maritime mondial, derrière les États-Unis et devant l'Australie. C'est une chance sur le plan économique, car cette économie représente aujourd'hui 14 % de notre PIB, mais c'est aussi une responsabilité importante lorsqu'il s'agit de la protection de la biodiversité, notamment marine.

la Chine, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam et la Thaïlande émettraient à eux seuls 6,5 millions de tonnes de déchets déversées dans les océans, dont une part d'ailleurs provient de nos propres pays.

total, plus de 10 000 projets sont menés dans 134 pays. Toutefois, ce dispositif est encore trop peu utilisé, car il est trop complexe pour les petites collectivités françaises. Dans le cadre de l'aide publique au développement, la France contribuera à hauteur de 1,5 milliard d'euros entre 2019 et 2023 pour alimenter le Fonds vert pour le climat. Ne devrait-on pas flécher une partie des investissements de ce fonds vers des projets permettant aux pays en développement de se doter de moyens pour mieux gérer ces déchets ? Nous aurons l'occasion d'en débattre lors de l'examen du projet de loi de programmation relative au développement solidaire pays s'est montré exemplaire depuis plusieurs années en permettant une prise de conscience généralisée de nos concitoyens et en adoptant des mesures ambitieuses pour protéger notre biodiversité et limiter la pollution par le La proposition de loi de notre collègue Angèle Préville, que je salue, ainsi que la rapporteure, s'inscrit dans la continuité de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite AGEC- je salue Marta de Cidrac -et fait écho au triste constat que je viens de dresser. La prise en compte de la pollution quasi invisible résultant des granulés ou des microbilles de plastique est une étape indispensable dans ce combat. Je ne peux que saluer cet engagement qui va dans le bon sens et qui est partagé par un grand nombre d'entre vous. Cependant, il reste beaucoup à faire. Cette proposition de loi est une étape. Je ne doute pas que le projet de loi Climat et résilience permettra de poursuivre les discussions sur ce sujet et d'apporter des réponses à traduire de façon pragmatique sur le plan législatif. Pour l'heure, le groupe Les Républicains votera ce texte.

de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, qui précise que, à compter du 1 janvier 2022, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels devront être dotés d'équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l'environnement.

qui a donné lieu à une consultation du public, reprendra le souhait qui a été exprimé en faveur d'un renforcement des mesures d'affichage. Je suis plus réservée quant à l'introduction d'une obligation de déclaration annuelle des pertes et fuites. C'est pourquoi ce projet de décret

leur emploi revient à déplacer le problème. Il n'existe pas aujourd'hui d'alternative écologique à ce type de recyclage de nos pneumatiques, qui permet d'économiser 60 % de CO2.

semble donc que nous brûlons les étapes. Troisièmement, les terrains synthétiques sont devenus un outil essentiel dans nos collectivités pour le développement du sport pour tous, car ils réduisent la pression d'usage sur les terrains engazonnés

À l'instar des ballons de baudruche, ces lanternes constituent une source de pollution. Une fois lâchées, elles deviennent des déchets qui se dispersent. Elles peuvent notamment comporter des parties métalliques. De plus, les risques d'incendie ne sont pas négligeables, puisque ces lanternes finissent toujours par retomber et peuvent s'accrocher à la végétation. Certaines préfectures ont donc adopté des arrêtés visant à interdire le lâcher de lanternes volantes en même temps que celui des ballons de baudruche. La mention « 100 % biodégradable » étant trompeuse, nous soutiendrons le sous-amendement de la rapporteure visant à supprimer la mention du caractère « non biodégradable » de ces lanternes volantes.

Mme la rapporteure. Cet amendement de précision rédactionnelle vise à s'assurer de l'application effective de l'article 3 en prévoyant qu'un lâcher de ballons soit assimilé à un abandon de déchets commis sur le lieu du lâcher. Cette précision facilitera l'exercice par le maire de son pouvoir de police.

Apposée sur le pare-brise des véhicules, cette vignette gratuite leur donnerait droit à une dérogation de circulation dans les zones à faibles émissions (ZFE). Ce texte a été cosigné par plus de quatre-vingts sénatrices et sénateurs. Je les en remercie chaleureusement. Pourquoi un tel engouement et pourquoi la nécessité d'un tel texte ? La pollution de l'air de nos grandes agglomérations étant de plus en plus importante, les ZFE sont à juste titre appelées à se multiplier. Ainsi, après Paris, le Grand Paris, Grenoble et Lyon, la loi d'orientation des mobilités a rendu obligatoire la création de ZFE dans sept autres métropoles : Aix-Marseille, Montpellier, Nice, Rouen, Strasbourg, Toulon et Toulouse. et résilience devrait encore accroître leur nombre. Elles vont donc concerner des dizaines de millions de nos concitoyens. L'objet de ces ZFE est de limiter la circulation des véhicules les plus polluants. pour circuler dans ces zones, les véhicules doivent avoir une vignette Crit'Air qui les classe selon leur niveau de pollution, les véhicules les plus polluants pouvant faire l'objet d'une interdiction de circuler. Comme l'a très bien rappelé la rapporteure, en commission, les véhicules de collection ne peuvent prétendre à une identification Crit'Air. Il revient aux intercommunalités de définir les règles de la ZFE,

La première est patrimoniale. Au même titre que les cathédrales, les gares et moult bâtiments publics et privés, les fleurons de notre industrie font partie intégrante de notre patrimoine. Quoi de plus symbolique de cette industrie que les véhicules anciens, qu'il s'agisse de tracteurs, de véhicules agricoles, militaires et de pompiers, de motos ou d'automobiles ? ? De la même manière qu'il faut entretenir notre patrimoine architectural, il faut entretenir ce patrimoine industriel. Dans cette conservation, l'usage et l'utilisation sont primordiaux. Pour les véhicules de collection, cela suppose de les faire rouler occasionnellement. La deuxième raison de ne pas abandonner les véhicules de collection est de nature économique. Cette filière, constituée principalement d'artisans et de très petites entreprises, compte 24 000 emplois dans plusieurs secteurs : la carrosserie, la mécanique, l'entretien, le négoce, l'événementiel, etc. etc. Son activité est croissante, avec un chiffre d'affaires annuel évalué à 4 milliards d'euros, soit le double de celui des sports mécaniques. À cela s'ajoute l'enjeu de la transmission des savoirs par l'apprentissage. argument fondamental, ces vieux véhicules que l'on voit de temps en temps parader dans nos rues et dans nos campagnes procurent de la joie et du bonheur non seulement à leurs propriétaires, mais aussi à tous ceux qui les admirent quand ils sont de sortie. À leur manière, ces vieux véhicules contribuent à renforcer le « vivre ensemble », le lien social et intergénérationnel si fragilisé en ces temps de crise sanitaire. Cette passion partagée n'a rien d'élitiste comme j'ai pu l'entendre dire. De nombreux véhicules de collection sont accessibles à des prix tout à fait modiques. Par exemple, une 4 CV Renault- qui fut d'ailleurs la première voiture française construite à plus d'un million d'exemplaires, mais surtout la première qu'un ouvrier pouvait acheter neuve -une 203 Peugeot ou une Simca Aronde peuvent être acquises pour quelques milliers d'euros.

: l'un de décentralisation, l'autre écologique et le troisième de légistique. Je vais répondre à chacun d'entre eux. Premièrement, mon texte serait en quelque sorte recentralisateur, puisqu'il créerait une possibilité nationale de dérogation aux ZFE pour les véhicules de collection. Si cela peut sembler vrai, il faut revenir au sens même de la décentralisation, à laquelle je demeure naturellement très attaché. La décentralisation et la différenciation qui en

le propriétaire d'une voiture ancienne puisse avoir le droit de circuler à Grenoble quand le propriétaire du même véhicule ne pourrait pas le faire à Lyon, sans aucune différence de situation La différenciation ne serait alors rien d'autre qu'une discrimination qui ne se justifierait pas. Autrement dit, bien défendre la différenciation, c'est la réclamer à bon escient

ils sont 20 000 fois moins abondants. Les véhicules de collection ont un impact extrêmement faible sur la qualité de l'air. l'air. L'Allemagne, que l'on ne peut pas soupçonner de laxisme environnemental, autorise la circulation de ces véhicules de collection dans les ZFE depuis plus de dix ans. Mes chers collègues, c'est ce modèle allemand, ni plus ni moins, que je vous propose de transposer en droit français, en adoptant ce texte. Il me reste à répondre à l'argument de légistique qui m'a valu l'avis défavorable de notre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, au motif que ce texte relèverait du règlement et non de la loi. Avec un peu de malice, je serais tenté de répondre que cette rigueur à défendre le domaine réglementaire n'anime pas souvent nos travaux. Combien de lois bavardes, aux articles éminemment réglementaires, n'avons-nous pas votées dans cet hémicycle ? ? Trêve de malice ! Le caractère réglementaire du présent texte n'est pas si évident que cela. Il découle du du fait que l'article de loi créant les ZFE renvoie à un décret la définition des catégories de véhicules dont la circulation dans une ZFE ne peut être interdite. C'est sans doute là que le bât blesse. Le législateur n'aurait pas dû abandonner ce point au pouvoir réglementaire, tout simplement parce qu'il touche à une liberté fondamentale, la liberté de circulation, la liberté d'aller et venir. venir. Dans cette proposition de loi, je propose au législateur de reprendre ses droits pour légiférer sur l'aménagement d'une liberté fondamentale. Je tiens à féliciter ma collègue Évelyne Perrot,

pour leurs millions de sympathisants, et pour continuer de voir briller les yeux des enfants quand le passé ressurgit dans nos rues et dans nos campagnes, sur deux, trois, quatre, et parfois même six ou huit roues ! La parole

durable. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant toute chose, je vous prie de bien vouloir excuser la rapporteure, Mme Évelyne Perrot,

non seulement aux 250 000 collectionneurs de voitures d'époque, mais aussi à des millions de sympathisants, aux territoires et aux élus qui organisent 6 000 à 7 000 manifestations par an, ainsi qu'à toute la filière « voitures de collection » qui représente, en 2020, grâce à son dynamisme, 24 000 emplois et 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le phénomène est encore plus profond. Avec beaucoup d'à-propos, un de nos collègues en commission a cité les travaux de Roland Barthes, qui dans les années 1960 plaçait la voiture dans la catégorie des mythologies françaises

sinon dans son usage, par un peuple entier qui s'approprie en elle un objet parfaitement magique. » Tout au long de ses travaux, la commission a été sensible à cette dimension qui semble appartenir au passé, mais dont nous témoignons qu'elle continue d'imprégner le présent et sans doute l'avenir. L'enjeu de cette proposition de loi qui vise à garantir la circulation des véhicules de collection tient à la préservation d'un double patrimoine, industriel et culturel. Un patrimoine industriel, tout d'abord : alors que nous souhaitons relocaliser l'industrie dans les territoires, il est essentiel de rappeler la place centrale des objets haut de gamme dans notre économie, avec parmi eux les véhicules d'époque. Le et l'excellence de fabrication sont autant de marqueurs de notre industrie automobile, dont les véhicules de collection sont en quelque sorte les porte-drapeaux. culturel, ensuite : les véhicules de collection procurent indéniablement des moments de convivialité dont notre pays a tant besoin Le passage de ces véhicules suscite l'enthousiasme et aussi l'apaisement dans les grandes agglomérations où la circulation est trop souvent crispée par des tensions entre les voitures, les deux roues, les trottinettes et les piétons. La passion intergénérationnelle suscitée par ces véhicules n'est d'ailleurs pas nécessairement liée à la richesse économique ni réservée aux très hauts salaires. Nous écartons le soupçon d'élitisme en rappelant la réalité : un véhicule de collection n'est pas nécessairement un véhicule très onéreux,

La proportion de motorisations diesel est, pour l'heure, très faible, ce qui évite la production de microparticules, mais la consommation d'essence des véhicules de collection est souvent plus élevée que la moyenne et s'accompagne donc de plus fortes émissions de CO2, tout particulièrement en cas de mauvais réglage, avec une très grande hétérogénéité en fonction de l'âge du véhicule. Néanmoins, tout élargissement du périmètre des véhicules d'époque aurait pour conséquence d'augmenter l'impact carbone de la circulation de ces véhicules. Alertée de l'existence d'une possible entrave à la circulation des véhicules de collection, la rapporteure a entendu plusieurs acteurs concernés par la mise en place des zones à faibles émissions.

Le ministère des transports a également confirmé que des discussions étaient en cours avec la Fédération française des véhicules d'époque pour inscrire les véhicules de collection parmi les dérogations nationales, au même titre que les véhicules de police ou de pompiers. Dès lors, la question qui nous est posée est de savoir si, au-delà du signal que nous envoyons, il nous faut voter une loi sur la libre circulation des voitures de collection. se prononcer en ce sens pour plusieurs raisons. Tout d'abord, dans les ZFE déjà mises en place, on n'identifie pas d'entrave à la liberté de circulation des voitures de collection. Ensuite, si par le passé, le Parlement a parfois légiféré dans le domaine réglementaire, nous sommes devenus plus exigeants. Je rappelle aussi que le Conseil d'État protège de façon systématique le domaine législatif et sanctionne les décrets qui s'aventurent dans le domaine de la loi. En l'occurrence, la loi renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les catégories de véhicules dont la circulation dans une ZFE ne peut être interdite. En fin de compte, si le législateur adoptait cette proposition de loi, il en résulterait une vraie dissymétrie avec, d'une part, une loi spécifique pour les voitures de collection et, d'autre part, un décret qui accorde des dérogations nationales pour tous les autres véhicules, voitures de police, de pompiers, etc. Je conclurai en rappelant deux éléments. Tout d'abord, la Fédération française des véhicules d'époque (FFVE) est venue au Sénat pour recommander de suivre le modèle allemand qui facilite la circulation de 595 000 véhicules de collection à travers les 85 zones écologiques allemandes. Or la transposition de cet exemple allemand passe nécessairement par la voie du décret. Il suffirait d'ajouter trois mots dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, très précisément à l'article R. 2213-1-0-1 qui « interdit d'interdire » l'accès à certains véhicules dans les zones à circulation restreinte. Ensuite et surtout, j'insiste sur le fait que le Sénat, grand conseil et protecteur des territoires, reste plus que jamais attentif à la nécessité de différencier les solutions locales ; or c'est très exactement la philosophie qui a présidé faibles émissions comme des outils à la disposition des collectivités territoriales. Jusqu'à maintenant, l'intelligence territoriale a fonctionné à plein régime en accordant aux voitures de collection la souplesse que nous préconisons. Rappelons qu'il ne s'agit pas là de la seule compétence de restriction de circulation dont sont dotés les maires, qui disposent d'autres pouvoirs portant sur la liberté de circulation. Notre commission a donc conclu l'examen de ce texte en adressant un message très positif pour la préservation d'un phénomène culturel, social et industriel. Toutefois, dans un souci de cohérence juridique avec nos travaux législatifs passés et à venir sur les ZFE, nous n'avons pas adopté le dispositif prévu dans cette proposition de loi, car il pourrait nous engager dans une mécanique juridique complexe. Surtout, faisons confiance à l'intelligence territoriale et évitons de susciter un raidissement de la part de ceux qui craignent qu'on ouvre la « boîte de Pandore » des dérogations législatives.

Les véhicules de collection sont une part de notre patrimoine, une tradition populaire, une trace de la place centrale qu'ont eue la France dans le développement de l'automobile et l'industrie automobile dans le développement de la France. Comme vous, le Gouvernement souhaite les préserver. Comme vous, le Gouvernement souhaite qu'ils puissent continuer de circuler. Nous sommes d'accord sur l'objectif ; il nous reste à nous accorder sur les modalités. Premièrement, votre texte pose le principe d'une dérogation nationale pour la circulation des véhicules de collection dans les zones à faibles émissions. Créées par la loi d'orientation des mobilités et renforcées par le projet de loi Climat et résilience, ces zones sont nécessaires pour améliorer la qualité de l'air dans les centres urbains les plus denses. C'est une question de santé publique. Vous craignez que leur mise en place dans plusieurs agglomérations françaises n'ait pour conséquence de limiter la circulation des véhicules de collection. Or ces derniers ne sont pas laissés sur le bord de la route : les ZFE mises en place ou en cours de l'être prévoient toutes, sans exception,

Actuellement, la seule dérogation nationale concerne les véhicules d'intervention, comme les camions de pompiers, les ambulances et les véhicules de police. Pour ces véhicules, nous ne pourrions en effet envisager qu'un délai pour la mise en place des dérogations empêche leur circulation,

Deuxièmement, votre texte vise à créer une « vignette » collection. Là encore, nous approuvons l'idée de mieux protéger les véhicules de collection, mais nous divergeons sur les modalités

Les critères actuels permettant d'obtenir la qualification de « véhicule de collection » ne sont pas assez restrictifs. Les normes européennes indiquent que tout véhicule de plus de 30 ans n'ayant pas été modifié peut y prétendre, en adressant une demande de « certificat collection » à la Fédération française des véhicules d'époque.

Le Gouvernement s'est attelé à définir des critères plus précis. Nous avons engagé un travail avec la Fédération française des véhicules d'époque en ce sens. Étant donné que ces véhicules sont plus anciens, ils sont aussi plus émetteurs au kilomètre parcouru, comme certains d'entre

exemple à restreindre l'âge des véhicules, pour n'accorder une dérogation qu'aux plus anciens, dont le caractère de collection semble pertinent ; à ne pas autoriser les trajets du quotidien pour ces véhicules, par exemple ceux entre le domicile et le lieu de travail ; à exclure de la dérogation certains types de véhicules plus polluants, comme les véhicules diesels ou les véhicules utilitaires ; à définir un kilométrage maximal annuel ; ou encore, à mettre en place un contrôle technique adapté pour assurer la sécurité de ces véhicules. Ces travaux embryonnaires doivent être poursuivis, et je suis très ouvert aux contributions du Parlement. Enfin et surtout, nous avons un troisième point de divergence, car tous les aspects de cette proposition de loi sont de nature réglementaire, tant la qualification des véhicules de collection que le niveau de dérogation aux ZFE. Il n'est donc pas nécessaire d'inscrire ces points dans la loi. Un décret en Conseil d'État suffira lorsque nous aurons trouvé sur les modalités d'application. Pour toutes ces raisons, et dans la lignée de l'avis que Mme la rapporteure a donné en commission, le Gouvernement ne soutient pas cette proposition de loi. Nous restons en revanche à disposition pour poursuivre le travail de qualification de ces véhicules avec la Fédération française des véhicules d'époque, et en lien étroit avec les parlementaires qui le souhaiteraient. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les amoureux de belles jantes et de carrosseries brillantes

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à n'en pas douter, si nous devions associer un siècle à un objet technologique, il n'y aurait rien de mieux pour caractériser le XX siècle que l'automobile, invention qui bouleversera la société, outil d'émancipation des individus qui favorisera la libération des mobilités. Il est intéressant de remarquer que le premier déplacement privé de plus de cent kilomètres en Allemagne a été effectué par Bertha Benz en 1888 : celle-ci utilisa l'invention de son mari pour aller, sans la permission des autorités, rendre visite à sa mère. L'automobile modifiera considérablement l'organisation du travail. Le taylorisme et le fordisme vont ainsi introduire le travail à la chaîne, l'hyperspécialisation des tâches, puis les flux tendus, les flux tendus, le et autres concepts poussant vers toujours plus de performance opérationnelle et d'optimisation des coûts. L'automobile est aussi l'une des caractéristiques de la puissance industrielle des États, qui sont souvent identifiés par les marques qu'ils produisent. C'est une industrie qui entraîne dans son sillage celle du pétrole qui marque, lui aussi, son siècle. Enfin, l'automobile a la capacité de façonner les imaginaires avec des compétitions en tout genre, des épopées et des sagas, mais aussi des représentations et un statut social. Roland Barthes ne s'y est pas trompé puisque, en 1957, dans son livre consacré aux mythes de la vie quotidienne française, il a consacré un article à la nouvelle DS. Hasard du calendrier parlementaire, y figure aussi un article sur ce nouveau matériau qu'est alors le plastique, symbole d'une forme de modernité qui, quelques décennies plus tard, aura colonisé notre planète. Le XX siècle s'est refermé sur le constat amer que notre modèle de développement touchait à ses limites. L'épuisement des ressources, le réchauffement climatique, la pollution de l'eau et de l'air nous poussent à nous interroger et à agir. C'est aussi dans ce contexte, celui d'un changement de paradigme, que nous devons analyser cette proposition de loi.

Certes, les véhicules de collection représentent une faible part des émissions de particules, mais, alors que les zones à faibles émissions mobilité (ZFEM) ont été créées pour protéger les populations contre la pollution issue du trafic routier, la qualité de l'air représente un enjeu majeur de santé publique. l'étude réalisée par Santé publique France, la pollution de l'air serait responsable de 48 000 décès prématurés par an en France. Le trafic routier est responsable de 57 % des émissions d'oxyde d'azote. Devons-nous ouvrir la voie législative à un contournement généralisé du dispositif, alors que d'autres solutions existent veut permettre à ces véhicules patrimoniaux de continuer à circuler ? À l'heure où les débats se concentrent sur le projet de loi Climat et résilience et la traduction législative des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, ne risquons-nous pas d'envoyer un message qui sera probablement mal perçu et susceptible d'être dénigré, et de déconsidérer notre institution ? La deuxième direction dans laquelle je vous propose d'avancer, c'est le domaine de la loi. Des dérogations générales à l'application du dispositif ZFE sont possibles. L'article R. 2213-1-0-1 du code général des collectivités territoriales dispose que l'accès à la zone de circulation restreinte ne peut être interdit aux véhicules d'intérêt général, aux véhicules du ministère de la défense, aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées, etc. Devons-nous compléter par voie législative cette liste de dérogations générales qui, elles, sont du domaine réglementaire ? Nos débats ont souvent illustré cette impérieuse nécessité de cantonner chacun dans son domaine respectif. Lors des débats de contrôle, combien de fois avons-nous dénoncé l'absence de publication

pour établir la liste des dérogations à la zone à faibles émissions mobilité pour les véhicules utilitaires légers et les poids lourds. Les véhicules de collection sont compris dans ces dérogations. C'est notamment le cas pour Grenoble-Alpes pour Grenoble-Alpes Métropole. N'oublions pas que le Sénat est l'assemblée des collectivités locales et que nous devons faire confiance au dialogue, à la compréhension mutuelle et à l'intelligence territoriale pour trouver les solutions adaptées permettant à ces véhicules de continuer à circuler. Sans sous-estimer la valeur patrimoniale des véhicules de collection, le poids économique représenté par ce secteur, le potentiel d'animation locale que représentent les manifestations et les rallyes, mais au vu des éléments développés, le groupe Socialiste, Écologiste

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

la passion des 250 000 collectionneurs qui rassemblent des centaines de milliers de véhicules et animent chaque année des milliers d'événements sur l'ensemble du territoire français, dont certains sont certes extrêmement prestigieux, mais dont l'immense majorité traduit

c'est de les voir fonctionner et, donc, de les faire circuler. Rien n'est plus triste pour ceux qui sont passionnés par ces

de ces véhicules n'ont pas la certitude de pouvoir rouler, c'est toute une filière qui sera remise en cause. À partir du moment où l'on ne trouvera plus d'artisans, d'ouvriers et de professionnels s'engageant, s'engageant, inquiets de leur avenir, à perpétuer ce savoir-faire, c'est peu à peu tout ce patrimoine qui s'étiolera et disparaîtra.

nous pourrions demain rencontrer des gens qui, à juste titre, se diront que ces véhicules n'ont simplement aucun intérêt, puisque nous n'aurons même plus la joie limitée,

qui se sont exprimés ici sont très favorables à ces témoignages du passé -, mais parce que, règlement après règlement, nous allons interdire de fait leur utilisation, sauf dans des conditions très exceptionnelles, en vertu d'autorisations préalables et sans doute de plans de circulation avalisés par des ingénieurs compétents, tous regroupés dans des comités d'approbation ... Il faut en rester à un principe de liberté.

Nous avons encadré ces évolutions dans la loi d'orientation des mobilités et étudierons de nouveau la question dans les discussions qui auront lieu ces prochains mois. Les voitures anciennes occupent une place toute particulière dans le coeur des Français. Environ un million de voitures anciennes sont en circulation sur notre territoire, ce qui représenterait 1,5 % du parc roulant. Les collectionneurs sont nombreux et passionnés C'est pourquoi je salue l'esprit du texte que nous examinons aujourd'hui, qui vise à la création d'une vignette « collection » pour les véhicules d'époque. Cependant, je comprends aussi les arguments avancés par M. le rapporteur et dont nous avons discuté en commission,

mais je reste persuadé que les solutions à l'échelon local sont plus pertinentes. Je suis également sensible à la problématique de la pollution de l'air, dont le trafic routier est l'un des grands responsables. Notre pays a d'ailleurs été condamné par la Cour de justice de l'Union européenne pour manquement aux obligations issues de la directive concernant la Cependant, les voitures anciennes ne représentent qu'une faible part de nos émissions : elles sont peu nombreuses et parcourent, chaque année, un kilométrage bien inférieur à la moyenne des véhicules en circulation en France. Leur impact est donc minime. minime. Il me paraît aujourd'hui crucial de préciser la définition et le cadre juridique des véhicules de collection. Il est essentiel d'ouvrir des discussions sur les conditions à remplir, afin de savoir où placer le curseur en la matière. Cela rendra l'identification de ces véhicules plus facile. J'aimerais également revenir sur les dérogations créées, d'abord en soulignant, comme beaucoup l'ont fait, que des dérogations locales sont déjà autorisées au niveau des ZFEM. Ces territoires ont tous accordé une dérogation aux voitures de collection. J'espère que les prochaines ZFEM feront de même. le monde du véhicule ancien est aussi un secteur économique important, avec des milliers d'emplois et un chiffre d'affaires de plusieurs milliards d'euros. Ce sont de nombreuses manifestations qui rassemblent des passionnés du monde entier.

C'est aussi l'histoire de fleurons industriels français, le cahier des charges de la Citroën 2 CV, ou encore l'évolution spectaculaire du de la DS. Les enjeux autour de la voiture sont aujourd'hui différents. Nous cherchons désormais à développer des infrastructures de mobilité qui s'éloignent de ce que l'on appelle le « tout-voiture ». Cette politique permettra de désenclaver les territoires ruraux et très peu denses, tout en luttant contre la pollution atmosphérique. des voitures plus propres. J'encourage bien sûr ces évolutions pour nos citoyens et nos territoires. Cependant, il suffit de voir les yeux pétillants des collectionneurs de voitures devant leur bolide pour comprendre les passions que suscite cette proposition de loi.

monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons un impératif : la lutte contre la pollution de l'air et ses conséquences sanitaires désastreuses. Les zones à faibles émissions (ZFE), les dispositifs de restriction de circulation des véhicules les plus polluants, sont donc des leviers nécessaires qui doivent être maniés de façon suffisamment ferme pour donner des résultats.

Oui, si l'on considère que l'intérêt général nécessite aussi la préservation de notre patrimoine et la pérennité des savoir-faire d'une filière artisanale de maintenance et de rénovation. si l'on considère que leur usage réel, quand il est raisonnable, en fait une source d'émissions marginales. En termes de santé publique et de qualité de l'air, leur interdiction n'améliorerait quasiment Comme alsacien, je connais un peu le fameux modèle allemand d'exemption : celui-ci est effectivement cohérent, pratique et donne satisfaction. Ce modèle nous montre qu'il est possible de bien cadrer, en jugulant les effets d'aubaine par une labellisation rigoureuse, rigoureuse, un dispositif permettant de concilier lutte contre les motorisations polluantes et maintien d'une culture populaire de préservation et d'usage récréatif des belles voitures d'autrefois. Cette proposition de loi va donc dans le bon sens. Le souci

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme la poule au pot sous Henri IV, l'automobile reste « un lieu de mémoire heureux dans l'imaginaire des Français Voilà comment l'historien des transports Mathieu Flonneau caractérisait, dans un entretien donné en 2019 au journal, le rapport des Français à l'automobile. Oui, nos concitoyens demeurent attachés à la culture automobile et à ce patrimoine historique qui nous ramène aux plus grandes heures de notre mémoire collective, qu'elles soient heureuses ou sombres. Rappelez-vous, mes chers collègues, ces célèbres tacots que furent les taxis de la Marne ou bien encore, dans un autre registre, le gang des tractions avant. L'automobile, même si elle est synonyme d'innovations permanentes, n'oublie pas pour autant son passé et ne manque jamais de célébrer ses ancêtres, avec un parc de véhicules de collection évalué à près de 300 000 dans notre pays. Souvent remises à neuf pour contrer les ravages du temps, bichonnées par leurs propriétaires qui y consacrent temps, moyens et énergie passionnée, ces véhicules forcent le respect, d'autant plus quand on les croise lors de leurs balades dominicales. La proposition loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans un moment particulier de notre histoire. La nécessité qui est la nôtre, qui doit être notre mantra collectif, est « d'aller à l'idéal et de comprendre le réel ». Nous savons toutes et tous que la transition écologique est une véritable priorité pour le bien-être collectif et même la survie de nos civilisations. Mais nous avons à relever le défi de la transition écologique ensemble : nous ne le relèverons pas les uns contre les autres, et encore moins les uns au détriment des autres. Voilà l'esprit qui doit nous animer lors de l'examen à venir du projet de loi Climat et résilience et de son article 27, qui fixe l'entrée en vigueur de zones à faibles émissions dans les agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants

Une disposition législative spécifique pour les voitures de collection n'est pas indispensable, car elle s'articulerait mal avec le cadre juridique existant en matière de déploiement des zones à faibles émissions mobilité. Notre débat a le mérite d'envoyer un signal positif au-delà de la seule communauté des propriétaires de véhicules de collection. En effet, nous voyons bien qu'il n'y a ni urgence ni péril. Bien au contraire, on assiste à un travail permanent de concertation et d'échanges entre les Monsieur le ministre, je vous sais très attaché à la concertation et au travail qui est conduit actuellement avec la Fédération française des véhicules d'époque. Comme l'a dit un jour Isaac Newton, « lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la pollution de l'air constitue un sujet préoccupant pour nos concitoyens qui en subissent les conséquences néfastes sur leur santé. Dans les grandes agglomérations françaises, les seuils d'exposition aux particules fines (PM2,5) dépassent les niveaux fixés par l'Union européenne, seuils qui sont eux-mêmes jugés insuffisants par l'Organisation mondiale de la santé Cette pollution a également un coût : une étude commandée par l'Alliance européenne de santé publique, fondée sur les analyses de la qualité de l'air de 432 villes européennes, évalue le coût de la pollution à 1 602 euros à Paris par an et par habitant, et à 1 134 euros à Lyon.

Conséquence de la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019, l'arrivée de nouvelles ZFEM ravive les inquiétudes légitimes des détenteurs de véhicules disposant de la carte grise « véhicule de collection » et de leurs admirateurs. Ainsi, sept nouvelles zones doivent être prochainement créées, tandis que le projet de loi Climat et résilience, actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, ajoutera les agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants d'ici à la fin de 2024, soit trente-trois zones supplémentaires.

a le mérite de ne pas ouvrir la voie à d'autres revendications intégrant les 900 000 véhicules dits « historiques » ou encore les, véhicules âgés de 20 ans à 30 ans, qui représentent environ 3 millions de véhicules. Toutefois, du groupe du RDSE suivra l'avis de la rapporteure. En effet, il n'y a pas d'urgence à légiférer. Au sein des quatre zones existantes, les véhicules de collection, en France ou ailleurs, conservent leurs prérogatives et ne subissent pas de mesures de restriction à la circulation. Laissons les collectivités territoriales concernées décider des modalités d'application de la loi et fixer les mesures qu'elles estiment les plus pertinentes pour améliorer la qualité de l'air des agglomérations. Les études d'impact qui précèdent les arrêtés de création d'une ZFE éclaireront cette décision et apporteront une réponse équilibrée et adaptée au territoire, en préservant sans doute la voiture de collection, comme dans l'ensemble des pays européens ayant institué de tels instruments, quelle que soit la tendance politique. Quelle tristesse de devoir troquer une traction avant, une Ford Mustang ou une Dodge Charger de collection contre une voiture électrique sans bruit et sans charme, d'autant plus que leur usage n'est pas identique. Certains producteurs d'automobiles ont l'intention d'électrifier des modèles mythiques, mais leur acquisition sera moins accessible. Mes chers collègues, la proposition de loi peut soulever des questions d'équité : une partie de nos concitoyens ne peuvent plus rouler avec des voitures considérées comme polluantes pour se rendre sur leur lieu de travail. Transports en commun saturés, voies de circulation encombrées où se multiplient les conflits d'usage, quelles alternatives leur offre-t-on pour se déplacer ? Lorsque la métropole du Grand Paris entend interdire la circulation des voitures thermiques d'ici à 2030, après le diesel en 2024, cela suppose d'écarter 99 % du parc automobile actuel en neuf ans. Malgré les diverses aides à l'achat cumulables, le reste à charge reste élevé. Dès lors, il ne nous apparaît pas opportun, d'un point de vue juridique et politique, de légiférer au profit de véhicules dont l'utilisation est restreinte à des usages non professionnels. Si le secteur du véhicule de collection devait être fragilisé dans l'avenir, envisager la publication d'un décret serait plus que souhaitable.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour commencer, je tiens à remercier notre collègue Jean-Pierre Moga d'avoir déposé cette proposition de loi que j'ai immédiatement cosignée. Cette dernière vise à créer une vignette « collection » donnant droit à une dérogation de circulation dans les Étant donné qu'une voiture de collection ne correspond à aucune catégorie du certificat qualité de l'air- Crit'Air -, le régime de circulation déjà dérogatoire doit être adapté, d'où l'intérêt de cette proposition de loi qui mérite néanmoins d'être contextualisée. Sur l'aspect « recentralisateur » de ce texte, je ne peux que souscrire aux propos de Jean-Pierre Moga. Bien qu'étant, comme beaucoup d'entre vous, un défenseur de la différenciation territoriale, il me semblerait incohérent qu'il y ait une liberté de circulation différenciée en fonction des territoires pour des véhicules qui, par définition, vont d'un point à un autre. vont d'un point à un autre. Cette liberté fondamentale ne doit pas s'apprécier exclusivement au niveau territorial, mais relève bel et bien du législateur. Il y va aussi d'une meilleure cohérence territoriale à laquelle je viens de faire allusion. Pour ce qui concerne l'argument écologique opposé à cette proposition de loi, il me semble qu'il doit être nuancé. Il est vrai que les moteurs d'antan et les émissions de gaz à effet de serre qui en découlent semblent, au premier abord, aller à l'encontre de l'impératif écologique sur lequel reposent toutes nos politiques publiques actuelles. En ce sens, la circulation de ce type de véhicules pourrait être considérée comme incompatible avec le développement des ZFE. Pourtant, l'opposition entre voitures anciennes et écologie ne nous paraît pas indépassable. La question que beaucoup se posent est de savoir si ces automobiles de collection, souvent décatalysées, et forcément plus polluantes, pèsent significativement dans la pollution globale en France. La réponse est non : leur part très minoritaire leur part très minoritaire dans le parc automobile français, leur utilisation occasionnelle, souvent à des fins de représentation, et leur circulation encadrée expliquent qu'elles ont une empreinte environnementale minime. Sur ce dernier point, l'usage non professionnel de ce type de véhicule doit être précisé : l'amendement déposé par Jean-Pierre Moga y contribue. En définitive, la Citroën DS, si chère à Charles de Gaulle-

Enfin, la dérogation accordée aux voitures de collection se justifie par la dimension culturelle et patrimoniale de ces véhicules. Le décret du 20 février 2017 relatif à la nomenclature des véhicules figurant à l'article R. 311-1 du code de la route et à la modification des règles relatives au contrôle technique des véhicules de collection précise qu'un véhicule de collection est un véhicule présentant un intérêt historique. l'ont rappelé : l'histoire de l'automobile, c'est un peu celle, non seulement de la chanson française, mais aussi du quotidien des Français. Des premières machines à vapeur aux prototypes à hydrogène, cette histoire témoigne tant du progrès technique que de l'évolution des modes de vie. de vie. Vous serez d'accord avec moi pour dire que la 2 CV, la Méhari, l'Alpine ou encore la Dauphine sont les témoins de leurs époques et de nos vies. L'utilité fonctionnelle d'une voiture se transforme au fil des décennies en valeur symbolique, donc patrimoniale. nos concitoyens vouent un véritable culte à ces reliques roulantes. Par exemple, le salon Retromobile, organisé chaque année à la porte de Versailles, a attiré en 2019 plus de 130 000 visiteurs en quelques jours. Une telle tendance est également perceptible dans les territoires.

Cette femme d'exception était en effet une pionnière de l'automobile féminine. Alors que le permis de conduire n'était pas nécessaire, elle avait obtenu, en 1898, une autorisation préfectorale pour conduire une voiture elle avait dû rapidement s'acquitter d'une amende de 5 francs pour « avoir circulé avec une vitesse exagérée dans le bois de Boulogne au risque de commettre un accident ».

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'automobile ancienne n'est pas réservée à une élite de collectionneurs fortunés, comme le rappelle une étude menée par les organisateurs du salon Retromobile qui fait référence en la matière. 250 000 familles, les membres de 5 000 clubs ou associations investissent leur temps libre, leurs économies et mettent en oeuvre une solidarité bienveillante pour partager, lors de près de 10 000 événements annuels, les bienfaits de ces liens sociaux qui nous font tellement défaut en cette période de crise sanitaire. En outre, 90 % des véhicules concernés sont ceux qui nourrissent l'imaginaire de la France d'après-guerre, celle des Trente Glorieuses : 4 CV, 2 CV, traction avant, DS, Ami 6, Renault 4, Peugeot 203, 403 ou 404 en sont les représentantes aux côtés de véhicules de marques étrangères ou de véhicules d'exception. Par ailleurs, cette filière, constituée principalement d'artisans et de très petites entreprises, compte plus de 20 000 emplois dans plusieurs secteurs d'activité de notre économie. Qu'il s'agisse de carrosserie, de mécanique, de négoce ou encore d'événementiel, cette activité est en croissance et son chiffre d'affaires annuel est évalué à 4 milliards d'euros. Sa préservation doit donc être encouragée, notamment au titre de sa singularité patrimoniale.

aux Français et ouvre la voie à de nombreuses autres dérogations. Je ne partage pas cette analyse. Les véhicules historiques représentent en effet moins de 2 % du parc de véhicules et 0,05 % des kilomètres parcourus. Ainsi, au regard des bénéfices tout à fait négligeables, voire indémontrables, qui en résulteraient pour la qualité de l'air dans les zones concernées, une interdiction ou des restrictions de circulation seraient totalement disproportionnées. En revanche, elles auraient des conséquences ravageuses pour de nombreux secteurs d'activité. Doit-on contraindre les propriétaires de véhicules de collection à ne plus se déplacer, même occasionnellement ? Les Français sont las de toutes ces interdictions. Ils veulent un peu de liberté Ils aspirent à une réelle qualité de vie et appellent de leurs voeux des mesures de préservation de l'environnement relevant du bon sens. Parce que ces voitures représentent une partie infime du parc roulant et que leur pollution est donc minime, je voterai, à titre personnel, en faveur de cette proposition de loi et, dès que je le pourrai, je m'achèterai une jolie voiture de collection ! La discussion

En outre, restreindre cette éligibilité aux seuls véhicules âgés de plus de quarante ans permet d'en exclure nombre de véhicules récents, plus polluants et présentant peu d'intérêt historique.

? Tout en reconnaissant l'importance des voitures de collection, la commission n'a pas adopté le dispositif de cette proposition de loi, pour des raisons juridiques et afin de laisser la main aux collectivités territoriales.

Bientôt, de nombreux véhicules vont entrer dans la catégorie réglementaire des véhicules de collection. Parmi eux, certains ne présentent que peu d'intérêt historique et sont, de surcroît, très polluants-

diesel : ce moteur à forte compression permet de tirer le meilleur parti d'un carburant pour un maximum de puissance. De plus, il a évolué dans le temps, et heureusement. Nous avons en Lorraine la plus grande usine européenne de fabrication de moteurs diesel.

Vous vous en doutez : je vous invite à ne pas suivre l'avis défavorable du Gouvernement et de la commission et donc à

il ne s'agit pas d'une fraude de pauvres et notre but n'est en aucun cas de stigmatiser les étrangers. Il s'agit d'une fraude en réseaux organisés, si bien organisés d'ailleurs que Tracfin, la cellule de renseignement financier

et enfin du rapport de la Cour des comptes. Cette proposition de loi a été consciencieusement examinée par les services du Sénat, que je tiens à remercier, pour éviter que des mesures réglementaires

Je maintiens, par exemple, que les conditions ne sont pas encore remplies, loin de là, pour éviter la fraude documentaire. J'attends avec impatience l'évaluation de l'article 13 du PLFSS portant consultation systématique par les organismes de sécurité sociale du fichier de Je maintiens également que la marge de progrès est très importante. Je sais que nos collègues du groupe communiste républicain citoyen et écologiste opposent la fraude fiscale à la fraude sociale

le Sénat a beaucoup travaillé sur la question de la fraude sociale ces dernières années. S'agissant de la commission des affaires sociales, je rappellerai ainsi le rapport de juin 2017 sur la lutte contre la fraude sociale de nos collègues Agnès Canayer et Anne Émery-Dumas mon rapport de juin 2019 sur la question plus circonscrite de la fraude à l'immatriculation à la sécurité sociale ; ou encore mon rapport de septembre 2020 à la suite d'une enquête commandée par la commission des affaires sociales à la Cour des comptes sur la fraude aux prestations de sécurité sociale. Nous avons également eu l'occasion de faire avancer la législation en matière de lutte contre la fraude lors de l'examen de plusieurs textes législatifs. Je pense en particulier à la loi de 2018 relative à la lutte contre la fraude, dont un volet est consacré à la fraude sociale,

et dans celui des organismes de sécurité sociale. Il s'agit de mettre en oeuvre les dispositions adoptées par le Parlement. Nous en attendons beaucoup, sachez-le. Je vous rappelle que l'un des amendements adoptés par le Sénat, qui n'a malheureusement pas été repris par l'Assemblée nationale, concernait la mise en oeuvre de dispositifs anti-fraude votés par le Parlement il y a dix et treize ans. Je note que, depuis lors, vous avez enfin pris les mesures d'application de l'un d'entre eux, qui concerne la procédure de déconventionnement d'urgence des professionnels de santé. le voeu, monsieur le ministre délégué, que le Gouvernement se montre bien plus diligent pour les mesures que nous avons adoptées cet automne. J'espère aussi que nous nous donnerons rapidement les moyens d'avoir enfin une vision claire et incontestable du dommage financier que représente la fraude, détectée ou non, pour chacun des régimes de sécurité sociale et dans tous les domaines : le recouvrement, les prescriptions et les prestations. (Mecss) m'a d'ailleurs missionné pour que je m'assure de la mise en place rapide des outils adéquats dans l'ensemble des caisses. C'est dans ce contexte que nous examinons aujourd'hui une proposition de loi de notre collègue Nathalie Goulet, dont nous connaissons l'engagement sur ce sujet.

au vu de la forte activité législative récente en matière de fraude, il a paru nécessaire à la commission de recentrer le texte, qui comptait initialement vingt-cinq articles, sur un nombre plus restreint de mesures clés.

Ainsi, chacun des articles qui demeurent porte sur un vrai sujet dont il est important que nous débattions en séance publique. Nous avons aussi maintenu ceux qui ne nous apparaissaient pas techniquement opérationnels afin que notre assemblée puisse décider en dernier ressort. Toutefois, comme je le disais en introduction, la qualité importe davantage que la quantité. Je voudrais ainsi mettre en avant plusieurs mesures de ce texte qui, aux yeux de la commission des affaires sociales, pourraient utilement renforcer nos moyens de lutte contre la fraude

En outre, cet article organise la transmission de ces informations entre les CAF et l'administration fiscale. Cela reprend des propositions formulées par la Cour des comptes dans l'enquête qu'elle nous a remise en septembre. Sur le fond, peut améliorer les contrôles, notamment de l'existence et de la conformité des logements donnant lieu aux versements d'APL. Il en va de même de l'article 14,

La commission a simplement souhaité recentrer cette avancée sur les prestations versées sous condition de résidence en France. Ces dispositions ne concerneraient donc pas les pensions de retraite, certains pensionnés vivant durablement hors de France et de l'Union européenne. L'article 15, que la commission a modifié en respectant l'intention de son auteur, auteur, permettra de renforcer les exigences que doivent satisfaire les pièces justificatives lors d'une inscription à la sécurité sociale ; à défaut, un entretien physique pourra être demandé de droit par l'organisme avant de procéder à l'inscription. Renforcer les exigences, c'est aussi apporter des moyens adéquats : nous ne pouvons pas entendre que certaines procédures sont insuffisamment sécurisées en raison du manque d'un scanner couleur, qui serait trop cher ! Même s'il risque de susciter des débats quant à la solution technique retenue, j'ai également à l'esprit l'article 17, relatif au domicile social des assurés sociaux. Mes travaux me conduisent à penser que le choix d'assimiler ce domicile social au domicile fiscal risque de poser des problèmes concrets à certains assurés. Néanmoins, cet article pose utilement la première pierre d'un chantier auquel, monsieur le ministre, j'espère que vous pourrez vous attaquer rapidement, au regard de l'utilité que pourrait présenter un tel domicile social en matière de calcul du juste droit et de lutte contre la fraude. ce texte a également entendu mettre l'accent sur la nécessité d'une meilleure coopération internationale en matière de fraude : nous partageons cette intention. Nous sommes convaincus, notamment, que la lutte contre les fraudes organisées passera par l'accélération et la systématisation des échanges au niveau européen. Enfin, je souhaite évoquer l'article 1, que nous avons supprimé et qui concernait le répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS). Je le rappelle, le RNCPS n'est pas une gigantesque base de données de la sécurité sociale, mais plutôt un portail ouvert aux organismes pour réaliser des requêtes essentiellement individuelles en faisant appel aux fichiers des caisses. C'est un sujet important sur lequel nous souhaitons aller plus loin dans les mois qui viennent à la lecture des conclusions de la mission que vous avez confiée à l'inspection générale des affaires sociales. Il est important, en effet, de faire évoluer cet outil. Nous devons avancer sur la question des systèmes d'information et des outils de gestion. Il y a là un enjeu de sécurisation du versement des prestations à bon droit, mais aussi un potentiel pour progresser en matière de réduction du non-recours aux prestations. Or je sais que nous sommes nombreux, sur ces travées, à vouloir améliorer l'accès aux droits. Telles sont, mes chers collègues, les principales conclusions de notre commission. Nous attendons avec impatience, monsieur le ministre délégué, que vous livriez votre analyse sur ce texte et que vous informiez le Sénat des principales mesures qui figurent dans la feuille de route que le Gouvernement compte adopter pour améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude sociale. La parole est à M.

Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Nathalie Goulet, lutter contre la fraude est une exigence fondamentalement démocratique, puisque c'est le corollaire de la nécessité d'une contribution commune telle que la prévoit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; cela permet aussi de rétablir l'équilibre entre les droits et les devoirs lorsque celui-ci est illégalement rompu. Les Français Les Français nous attendent, légitimement, sur ce sujet. Nous devons répondre à cette attente en considérant que la lutte contre la fraude est une obligation de principe qui s'impose d'autant plus quand les moyens engagés sont d'une ampleur inédite, comme c'est le cas durant cette période.

liminaire, sur la notion d'équilibre, sur la volonté de dépassionner le débat et de s'attaquer à la fraude aux cotisations comme aux prestations, en rappelant les ordres de grandeur et l'importance de la première par rapport à la seconde. Je veux aussi mettre à profit cette séance pour rappeler les progrès qui ont été faits en la matière. De nombreux rapports ont récemment souligné les améliorations déjà apportées au cours des dernières années, notamment sur la forte dynamique en volume et en montant de la fraude aux prestations détectée et sanctionnée, en augmentation de 30 % en un an, soit un niveau trois fois supérieur à celui d'il y a dix ans. Il faut aussi souligner la professionnalisation croissante de la lutte contre la fraude aux prestations comme aux cotisations, temps plein directement affectés à cette mission au sein des caisses, avec un meilleur ciblage des contrôles et des échanges d'informations croissants avec d'autres administrations et organismes. Tous ces rapports, au premier rang desquels celui de la sénatrice Nathalie Goulet et de sa collègue, la députée Carole Grandjean, ont inspiré cette proposition de loi, ils ont également souligné le travail qui reste à effectuer et ont appelé les organismes de sécurité sociale

Je souhaite aussi profiter de l'examen de cette proposition de loi pour vous donner trois illustrations concrètes de l'engagement du Gouvernement dans la lutte contre la fraude sociale. Tout d'abord, dans le cadre de l'examen de la dernière loi de financement de la sécurité sociale,

de la biométrie ; l'expérimentation prévue cette année va permettre d'ouvrir une nouvelle possibilité de sécurisation du versement des pensions, tout en allégeant les contraintes administratives qui pèsent sur les assurés. Dans le cadre du plan de lutte contre la fraude que j'ai eu l'occasion de présenter le 2 février, nous avons prévu des moyens humains pour procéder à un certain nombre de contrôles sur place, de manière à être plus efficaces dans le recensement et la détection de ce type de fraude. sociale pour 2021 prévoit de renforcer les contrôles et les sanctions des professionnels de santé, avec une obligation d'inscription à l'ordre et un déconventionnement d'office pour les professionnels condamnés pour fraude pour la seconde fois en cinq ans. Ce texte prévoit aussi des mesures permettant le renforcement des sanctions en cas de non-signalement d'un changement de situation, ou encore un doublement des plafonds de pénalité, à la main des directeurs des branches vieillesse Par ailleurs, Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé, et moi-même veillerons- vous avez dit, monsieur le rapporteur général, madame la sénatrice, votre attention sur ce point -à ce que la mission d'inspection qui aurait dû remettre son rapport parlementaire sur le répertoire national commun de protection sociale en 2020 puisse le faire avant la fin du premier semestre de cette année, le retard ayant été très largement enregistré pendant les périodes de confinement. L'objectif est de nous permettre de mieux cerner les usages de cet outil de partage des informations en temps réel entre les différents organismes qui interviennent dans le champ de la protection sociale. La mission doit notamment nous éclairer sur les usages actuels de ce répertoire en étudiant la possibilité et l'utilité d'avoir accès à des informations non encore mutualisées. J'ai également demandé

Enfin, j'ai demandé en décembre 2020, toujours avec le ministre des solidarités et de la santé, mais aussi avec la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, au directeur de la sécurité sociale de piloter le plan d'action, de prévention et de lutte contre la fraude sociale que j'ai présenté lors du premier comité de pilotage le 2 février dernier. Ce plan a vocation à décliner opérationnellement les mesures dont nous avons discuté avec vous et que nous allons de nouveau évoquer cet après-midi. Validé et partagé par tous les acteurs, il nous permet de mieux coordonner et de structurer notre politique de lutte contre la fraude.

Je ne considère pas que cette étape de travail- l'application des dispositions prévues en loi de financement de la sécurité sociale et la mise en oeuvre de ce plan de lutte contre la fraude -soit un aboutissement, c'est le début d'une démarche de renforcement de la lutte contre la fraude qui doit aboutir à un vrai changement d'échelle ce plan sera, au fil de nos échanges, renforcé, actualisé et enrichi. Je suis évidemment disposé, par construction et en application du droit, mais aussi par respect du Parlement, à faire réaliser toutes les évaluations que vous avez évoquées que vous avez évoquées dans les meilleurs délais et à m'assurer que l'ensemble des parlementaires des commissions concernées au Parlement soient régulièrement informés, autant qu'ils le souhaiteront, de la mise en oeuvre de ce plan et de son évaluation. Vous verrez ainsi que nous partageons les mêmes préoccupations et les points d'attention qui ont donné lieu à la rédaction de cette proposition de loi, même si certaines des mesures que celle-ci contient ne nous semblent pas nécessairement applicables immédiatement ou en l'état.

de ces risques ; la sécurisation des processus d'immatriculation et d'identification des assurés en généralisant le procédé d'attribution du numéro d'identification par un numéro d'attente, pour les réseaux qui ne l'appliquaient pas encore ; la sécurisation, de même, du processus de contrôle de l'existence à l'étranger- nous y reviendrons dans nos échanges, j'ai évoqué les moyens humains que nous allons mettre en place

plan contient, enfin, des mesures sur la maîtrise de la fraude aux cotisations et aux prestations de service internationales, sujet sur lequel l'information du Parlement pourrait encore être renforcée. Je serai particulièrement attentif à ce qu'un suivi précis, avec des actions concrètes et quantifiées, ainsi que des indicateurs permettant d'évaluer fidèlement l'atteinte des objectifs et que cela se traduise dans les nouvelles conventions d'objectifs et de gestion qui seront signées avec les organismes de sécurité sociale. Je veux dire notre attention et le soutien que nous apportons tout particulièrement à deux articles de la proposition de loi.

Les autres dispositions nous posent certaines difficultés, parce que nous portons une appréciation sur leur opportunité, parce que nous considérons qu'elles seraient difficilement applicables ou encore parce que nous avons fait le choix d'y donner suite différemment. Nous devons collectivement nous fixer une obligation de moyens, mais aussi de résultats et faire connaître le bilan de nos actions. Le débat qui va commencer est une manière de le faire et j'en remercie de nouveau l'auteure de la proposition de loi, tout comme je remercie, par avance,

les contournements des règles, les dissimulations et les détournements de recettes qui doivent être affectées aux régimes de sécurité sociale, mais aussi de contribuer à une meilleure efficacité et donc à une plus grande solidarité de l'ensemble de notre système de protection sociale. En cela, le débat qui s'ouvre est nécessairement utile. La parole est

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi tendant à appliquer vingt-quatre mesures urgentes pour lutter contre les fraudes sociales, présentée par Mme Nathalie Goulet, s'inscrit dans la longue liste d'initiatives récentes de la majorité sénatoriale contre la fraude sociale, sans compter les multiples amendements aux deux derniers projets de loi de financement de la sécurité sociale déposés par l'auteure de la présente proposition de loi.

qui insiste sur le fait que l'intensification de la lutte contre la fraude sociale est source d'atteintes aux droits des usagers ; qui pointe le fait qu'un « allocataire ou assuré de bonne foi, même s'il demeure responsable de son erreur ou de son oubli, ne saurait être qualifié de fraudeur et se voir appliquer des sanctions

ces pouvoirs sont d'autant plus dévastateurs que des ménages se trouvent dans l'obligation de procéder à des remboursements d'indus considérables au regard du budget du foyer, aboutissant à un affaissement des ressources de certains foyers au sein d'une population déjà fragilisée et qui, parfois, ignore ses droits. Cela confirme les résultats d'une enquête du même Défenseur des droits, publiée en mars 2017, qui révélait que les personnes en situation de précarité économique et/ou sociale rapportent plus de difficultés pour résoudre un problème avec une administration ou un service public, et qu'elles sont plus susceptibles d'abandonner leurs démarches.

complémentaire (CMU-C) et entre 53 % et 67 % pour l'aide au paiement de la complémentaire santé (ACS). Quant aux aides à la famille, une autre étude de 2018 estimait qu'entre 7,5 % et 8,2 % des allocataires ne recourent pas à leurs droits. Les principales raisons proposées pour expliquer que certaines personnes se retrouvent dans des situations de non-recours sont le manque d'information et la lourdeur administrative. Cela soulève notamment l'enjeu du risque de pauvreté et de l'approfondissement de la précarité sociale. Des enquêtes ont en effet montré que le recours au RSA n'est pas systématique, en raison, principalement, de la méconnaissance de ce dispositif. Ce problème se décline sur tous les secteurs de la protection sociale. Par exemple, pour le risque vieillesse, à l'âge de 70 ans, 32 % des assurés des régimes de retraite français nés en 1942 n'ont pas demandé tout ou partie de leurs pensions de retraite. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat estime que, si l'on peut juger que la lutte contre la fraude concernant les droits des usagers du service public est une politique publique légitime, celle-ci doit être équilibrée. Il se trouve que la fraude aux prestations sociales est bien moins importante que le non-recours aux droits. Il faut rappeler ici que, en 2015, la fraude aux prestations sociales représentait 673 millions d'euros, contre 4 milliards d'euros pour le non-recours au RSA. Ce n'est, bien évidemment, pas une raison pour ne pas lutter contre ces agissements. Il demeure néanmoins que les initiatives législatives sont bien plus fréquentes en faveur de la lutte contre la fraude que contre le non-recours, notamment de la part de la majorité sénatoriale. Les dispositifs de plus en plus étoffés de lutte contre la fraude laissent par ailleurs accroire à une fraude massive des bénéficiaires. Ce n'est évidemment pas le cas, mais cela traduit une vision tronquée de la situation. Ce sont 0,36 % des allocataires de la CNAF qui frauderaient délibérément, en revanche, 75,5 % des « fraudes » sont en fait dues à des omissions ou à de fausses déclarations, 16,5 % sont des fraudes à l'isolement et 8 % sont des faux et usages de faux. contre la fraude entretient donc la recherche de boucs émissaires, la dénonciation de l'assistanat et conduit, en creux, à une remise en cause de notre modèle social. Certains discours sur la fraude sociale tendent, en outre, à entretenir volontairement le flou entre la fraude organisée des réseaux, qui relève de la délinquance, et celle des individus isolés, bien plus facile à stopper. Par ailleurs, les bénéficiaires des prestations ne sont pas forcément les plus fraudeurs. Ainsi, pour l'assurance maladie, 47,5 % du montant des fraudes et fautes détectées relèvent des professionnels de santé, 31,1 % des établissements, 21,1 % des assurés et employeurs. À la demande de la commission des affaires sociales du Sénat, la Cour des comptes a estimé les préjudices des principaux organismes sociaux en 2019 à 1 milliard d'euros. Ce montant doit être mis en regard des 5,6 milliards d'euros de fraude fiscale recouvrés par l'État en 2018. La fraude sociale, y compris celle qui n'est pas détectée, est évaluée entre 14 et 45 milliards d'euros, alors que la fraude fiscale est estimée entre 66 et 88 milliards d'euros, voire 100 milliards d'euros pour certains syndicats des finances publiques. Cela suggère qu'il pourrait être nécessaire de hiérarchiser les priorités. Nous ne sommes cependant pas naïfs, nous savons bien que les différentes fraudes existent, mais nous ne souhaitons pas voter une proposition de loi qui laisserait accroire que cette fraude aux allocations sociales serait devenue un sport national. Nous appelons plutôt à une amélioration des dispositifs d'aide sociale qui permettrait de limiter la possibilité de fraudes. Nous souhaitons donc que soient mis en parallèle les moyens dévolus à la lutte contre la fraude sociale et les moyens déployés pour la lutte contre le non-recours,

nous entamons aujourd'hui l'examen en séance de la proposition de loi tendant à lutter contre les fraudes sociales. Je tiens, tout d'abord, à saluer le travail effectué par notre collègue Nathalie Goulet, auteur du texte, et par le rapporteur Jean-Marie Vanlerenberghe. Néanmoins, je forme également le voeu que nous puissions travailler à l'avenir sur un texte visant à lutter contre tous les types de fraudes, car chaque fraude est un coup de poignard porté à notre idéal républicain et le symptôme d'une société qui se détourne progressivement de l'intérêt collectif au profit des intérêts particuliers. La lutte contre les fraudes sociales est un sujet qui revient de manière récurrente sur les bancs de cette assemblée. Pour ne citer que les travaux récents, nous pouvons évoquer la proposition de résolution visant à lutter contre la fraude transfrontalière, déposée par notre collègue André Reichardt et votée par le Sénat, ou encore la proposition de loi tendant à instituer une carte vitale biométrique, déposée par notre collègue Philippe Mouiller et dont la présidente Catherine Deroche a été rapporteure. Notons également qu'une commission d'enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales, présidée par notre collègue député Patrick Hetzel, a été mise en place à l'Assemblée nationale. Ses conclusions ont été présentées en septembre dernier. Enfin, je rappelle qu'une proposition de loi visant à améliorer l'accès aux droits et à lutter contre la fraude sociale, déposée par notre ancien collègue Éric Doligé et dont j'étais la rapporteure, avait été discutée en mai 2016 au sein de cet hémicycle.

À ce titre, j'ai déposé plusieurs amendements inspirés de mon rapport sur la proposition de loi Doligé, visant à compléter les différents dispositifs présents dans la proposition de loi discutée ce jour. Les chiffres en matière de fraudes sociales divergent, mais je n'entrerai pas dans ce débat, car bien malin est celui qui peut se targuer de mesurer objectivement le montant total de ce type de fraudes. Le RSA, les aides au logement, les allocations familiales, le minimum vieillesse, les arrêts maladie sont autant de dispositifs concernés par ce phénomène en augmentation permanente. Quelques chiffres, tout de même, ont pu être vérifiés et sont symptomatiques des défaillances de notre pays à endiguer cette terrible réalité : il y a près de 74 millions de personnes bénéficiaires de prestations sociales, dans un pays qui compte 67 millions d'habitants plus de 250 porteurs de la carte Vitale ont plus de 120 ans et plus de 3 millions d'entre eux sont centenaires, voilà qui pourrait faire pâlir le Japon, champion de la longévité et qui aurait pu inquiéter Jeanne Calment dont le record tenait jusqu'alors L'enquête sur la fraude aux prestations sociales réalisée par la Cour des comptes à la demande de la commission des affaires sociales du Sénat et présentée en septembre 2020 permet de constater « qu'il s'agit bien d'une atteinte au principe de solidarité et d'un coût financier élevé Le Conseil constitutionnel a lui-même reconnu à la lutte contre la fraude le caractère d'une exigence constitutionnelle. Ne nous trompons pas, il s'agit bien ici de lutter contre la fraude organisée. un an de la prochaine élection présidentielle, il faut du courage politique, monsieur le ministre, pour s'attaquer à ce problème épineux et complexe. J'espère que l'exécutif est prêt à assumer ce courage. De nombreuses solutions existent et ne demandent qu'à être mises en place. Ce ne serait que justice, pour la majorité de nos compatriotes, silencieux par pudeur et honnêtes par valeur, ces femmes et ces hommes qui, chaque jour, font honneur à cette nation en se demandant ce qu'ils peuvent faire pour leur pays, et non l'inverse, conformément à la célèbre maxime du président Je ne sais si ce texte sera inscrit prochainement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, mais il a le mérite de remettre sur la table cette réalité qui n'est pas digne de notre pays et qui est une offense aux pères fondateurs de la sécurité sociale et aux personnalités politiques qui ont oeuvré et oeuvrent encore chaque jour en faveur de la solidarité nationale, pour que les plus faibles puissent être accompagnés par la puissance publique. La parole

De surcroît, même la Cour des comptes, dans son rapport présenté en septembre dernier, s'est estimée incapable de chiffrer avec précision ces pratiques. Tout indique pourtant que les montants des fraudes aux prestations et aux cotisations ont largement augmenté ces dernières années. À titre d'exemple, le montant de la fraude aux organismes sociaux est estimé par la Cour des comptes à 1 milliard d'euros en 2019, contre 850 millions d'euros en 2017. De plus, on dénombre près de 3 millions de bénéficiaires « fantômes » de droits à l'assurance maladie : c'est absolument considérable ! La fraude fait peser le doute sur l'efficacité et sur l'équité de notre modèle social. Il faut le constater : aujourd'hui, nos organismes sociaux ne sont pas assez armés pour lutter contre la fraude tant des particuliers que des professionnels. Aussi, nous devons urgemment nous atteler à repenser l'architecture de nos bases de données. Je pense notamment au répertoire national commun de la protection sociale. La principale difficulté réside dans le fait que toutes les prestations sont versées sur une base déclarative, avec un contrôle. Il faut travailler au croisement des données entre les organismes sociaux et fiscaux, il faut aussi leur donner accès aux historiques des montants versés afin d'éviter les doublons. Les moyens technologiques actuels doivent nous y aider. C'est dans cette même logique que je soutiens le développement de la carte biométrique : elle doit être totalement sécurisée. D'ailleurs, l'expérimentation actuelle doit rapidement laisser place à sa généralisation.

Il n'est pas acceptable, dans un pays aussi développé que le nôtre, avec un système aussi généreux que le nôtre, que nous ne disposions pas de moyens de contrôle plus performants. Pour conclure, mes chers collègues, la pérennité de notre modèle social dépend de notre capacité à lutter contre ces fraudes. Par conséquent, vous l'aurez compris, le groupe Les Indépendants soutient cette proposition de loi qui va clairement dans le bon sens. Il est temps d'agir. Il y va de la crédibilité de l'État, de la puissance publique et de l'avenir de notre modèle social. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la crise sanitaire qui dure se transforme de plus en plus en crise sociale et humanitaire, partout dans le monde. En France, 10 millions de personnes vivent désormais sous le seuil de pauvreté. L'Insee relate que la situation financière des ménages s'est fortement dégradée, avec une perte de près de 3 % des revenus, ce qui ne s'était pas produit depuis 1949. Par ailleurs, près de 700 000 emplois ont disparu en 2020, majoritairement des emplois à destination des personnes en situation de précarité. Pourtant, dans ce contexte, alors que la pauvreté s'étend et touche de nouveaux publics, alors que 20 % des ménages les plus pauvres ont dû massivement désépargner le peu d'économies qu'ils avaient pour faire face aux dépenses incompressibles, ce qui présage d'effets sociaux dramatiques partiellement différés par cet amortisseur, et alors que les associations nous enjoignent, pour prévenir ce phénomène, de lutter contre le non-recours aux droits sociaux et d'améliorer l'accès aux droits, notamment des plus jeunes, les mesures urgentes dont nous débattons aujourd'hui concernent la lutte contre la fraude sociale. Tout comme pour la réforme de l'assurance chômage du Gouvernement, il est difficile d'être plus anachronique, plus décalé par rapport à la situation sociale et plus déséquilibré ! En effet, alors que la fraude sociale concerne quasi uniquement ici

Cela s'explique par la focalisation constante, en raison des déficits sociaux, sur les seules dépenses sociales, qui sont scrutées avec attention, alors que les manques à gagner en recettes dus à la fraude ou aux optimisations de toute sorte sont quasi ignorés. Or le solde résulte bien des deux. la lutte contre les différentes fraudes est légitime, ce parti pris ne l'est pas. Le texte concentre notre attention sur la fraude aux prestations, y compris par des articles déjà satisfaits par le droit en vigueur. nombreux articles visaient à accroître les moyens de contrôle, mais surtout de surveillance des bénéficiaires des aides sociales, au mépris du respect de leur vie privée, comme si on les soupçonnait d'être, par nature,

le croisement des données à l'automatisation des droits, plutôt que de n'en envisager l'usage qu'au service du contrôle ? Nulle justification à la surveillance des données internet, comme le propose l'article 4, ou à donner des pouvoirs judiciaires aux organismes de sécurité sociale, comme le suggère l'article 18. La priorité de notre temps législatif doit être la lutte contre la paupérisation en cours et le renforcement de notre système d'aides sociales. C'est ce que la crise que nous vivons requiert et nous demande ! En conséquence, le groupe GEST votera contre

la proposition de loi de notre collègue Nathalie Goulet tend à s'attaquer à la fraude sociale une série de mesures, vingt-quatre avant son examen en commission des affaires sociales. J'y reviendrai dans quelques instants. Ces dernières années, des rapports et des enquêtes ont permis de mieux comprendre l'ampleur de la fraude sociale dans notre pays et d'y faire face plus efficacement. Il y a bien sûr le rapport de mission que vous avez rédigé avec la députée Carole Grandjean au mois d'octobre 2019, Goulet, à la suite duquel un important travail de fiabilisation du parc de cartes Vitale a été mené. Au Sénat, la lutte contre la fraude a été au coeur des travaux de la commission des affaires sociales. Au mois

de septembre 2020, une communication de la Cour des comptes révélait par ailleurs que le préjudice subi ou évité, au titre des fraudes avérées ou suspectées, s'élevait à 1 milliard d'euros en 2019. Ce sont près de 290 millions d'euros pour l'assurance maladie, soit 1,8 fois plus qu'en 2010. Face à ce constat, que peut faire le législateur et qu'a-t-il déjà fait ? Des mesures visant à lutter contre la fraude sociale ont été récemment votées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Je pense notamment à l'annulation automatique du numéro de sécurité sociale obtenu frauduleusement, au conditionnement des remboursements de l'assurance maladie aux professionnels de santé à leur inscription à l'ordre dont ils dépendent ou encore au déconventionnement des professionnels de santé condamnés à plusieurs reprises pour fraude. Ces mesures, dont certaines n'ont pas encore produit leurs effets, doivent faciliter le travail des 4 300 agents qui oeuvrent quotidiennement au sein des réseaux des caisses de sécurité sociale. C'est d'ailleurs dans cette optique que le Gouvernement a récemment créé une mission interministérielle de coordination anti-fraude, la Micaf. La proposition de loi de Nathalie Goulet s'inscrit dans cet esprit et tend à aller plus loin et plus vite. Si certaines mesures nous semblent intéressantes- c'est le cas notamment de l'article 15 qui exige une copie en couleur du titre d'identité pour l'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques -, d'autres nous paraissent en revanche prématurées, voire déjà satisfaites. C'est le cas de l'article 10 qui tend à sécuriser les données des certificats de vie des conventions avec des organismes de retraite d'États étrangers. C'est également le cas de l'article 21, déjà satisfait, qui supprime le conventionnement des professionnels de santé en cas de fraude manifeste. Mes chers collègues, la lutte contre la fraude sociale est évidemment une priorité, mais elle ne peut se faire que par étapes, afin d'assurer son efficacité et sa lisibilité par ceux qui en ont la charge. Si nous ne sommes pas opposés à l'esprit de ce texte, il nous semble donc préférable, compte tenu des différents éléments évoqués, d'attendre que les mesures adoptées ou mises en oeuvre ces dernières années fassent leurs preuves, afin de ne pas

La fraude remet en cause ce principe et doit donc, à ce titre, être combattue. Cette proposition de loi, déposée par Nathalie Goulet, semble avoir suscité quelques débats au sein de la commission des affaires sociales. J'entends les arguments avancés par certains de nos collègues qui dénoncent une stigmatisation. la fraude sociale n'est pas « la fraude des pauvres ». Elle est le fait d'un public très hétérogène qui ne manque ni d'idées ni de moyens, comme l'a relevé la Cour des comptes. Très bien ! Face aux difficultés rencontrées actuellement par des millions de nos concitoyens, la fraude, qu'elle soit fiscale ou sociale, est inacceptable. Depuis plusieurs années, les rapports pointant les faiblesses en matière de lutte contre la fraude sociale se multiplient. Au mois de septembre dernier, la Cour des comptes estimait que les progrès étaient encore bien trop lents. où les finances publiques sont fortement éprouvées par la crise sanitaire, lutter contre la fraude doit permettre une meilleure justice sociale. Comme l'a déjà rappelé l'auteur de la proposition de loi, « il faut que l'argent aille vraiment là où les gens en ont besoin Si la fraude aux prestations et cotisations sociales détectée en 2019 s'élève à 1,5 milliard d'euros, nous savons qu'elle est en réalité beaucoup plus élevée. Il est malgré tout extrêmement difficile d'en évaluer l'ampleur et les chiffres sont l'objet de fantasmes et de controverses. Selon l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la fraude aux cotisations sociales représenterait un manque à gagner de 7 à 9 milliards d'euros. aux prestations sociales, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale l'a récemment estimée à 14 milliards d'euros, certains parlant même de 30 milliards d'euros. La question qui se pose aujourd'hui est donc bien de savoir quels moyens nous pouvons mettre en place pour la combattre. Cela a été dit : cette proposition de loi est perfectible. Pour autant, sur un sujet aussi complexe, la rédaction issue des travaux de la commission des affaires sociales me semble amorcer une première étape. Certaines dispositions vont dans le bon sens. Je pense à l'obligation du versement des prestations sociales sur un compte français ou européen, à l'obligation de fournir des documents de bonne qualité pour les ressortissants étrangers demandant un numéro de sécurité sociale ou encore à la volonté de soumettre les dirigeants d'entreprises éphémères à des obligations déclaratives renforcées. Je me félicite également que le rapporteur ait proposé qu'un certain nombre d'articles soient maintenus pour permettre un débat avec le Gouvernement. C'est toujours à l'honneur du Sénat de chercher à prolonger le dialogue et de poser ainsi les jalons de nos prochaines réflexions. Souhaitons que le travail se poursuive également avec le plan que vous avez validé au début du mois de février dernier, monsieur le ministre, et qui comporte une trentaine d'actions. Il faudra également que nous nous penchions sur la question du non-recours. Selon les chercheurs de l'Observatoire des non-recours aux droits et services, chaque année, des milliards d'euros de prestations ne sont pas réclamés par des personnes qui y auraient pourtant droit. Cela s'explique notamment par la complexité de la législation et des démarches.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer l'opiniâtreté dont fait preuve notre collègue Nathalie Goulet dans son combat contre la fraude. Nous partageons d'ailleurs avec elle l'idée que la fraude remet en cause le consentement à l'impôt, pilier de notre société. En revanche, nous refusons de pointer du doigt les bénéficiaires des prestations sociales comme les principaux fraudeurs. Tant en nombre qu'en montant, les allocations familiales représentent une part minoritaire des fraudes qualifiées. Surtout, ces fraudes sont pour 70 % des omissions.

Pour nous, les vrais fraudeurs ce sont les 15 000 Français ou entreprises tricolores qui sont établis au Luxembourg et qui soustraient à l'impôt 6 500 milliards d'euros Les fraudeurs, ce sont les 166 filiales d'entreprises du CAC 40 qui détiennent des avoirs au Luxembourg. Ce sont les 80 milliards d'euros de fraude fiscale, c'est-à-dire de pertes de recettes pour le budget de l'État. Les fraudeurs, ce sont aussi les patrons qui ne cotisent pas à la sécurité sociale et qui, chaque année, font perdre 8 milliards d'euros à l'hôpital et à notre régime de retraite. Malheureusement, cette proposition de loi ne s'attaque absolument pas à cette fraude. Vous préférez pointer du doigt la fraude aux prestations sociales. Nous pensons que cela stigmatise les pauvres. Vous pointez du doigt les petits tricheurs qui cachent les grands voleurs Cette fraude aux prestations sociales est chiffrée par la Cour des comptes à 1,2 milliard d'euros, qu'il faut mettre en regard des 450 milliards d'euros de prestations versées par la sécurité sociale, soit moins de 0,3 % du total. Concernant la fraude documentaire, elle serait située entre 117 millions d'euros et 138 millions d'euros, bien loin des 14 milliards d'euros évoqués par certains. Contrairement aux idées reçues, en 2019, les fraudeurs ne sont pas celles et ceux que l'on croit. Ainsi, la fraude à l'assurance maladie provient, dans seulement 21 % des cas, des salariés

En comparaison, le non-recours aux prestations sociales atteint un montant largement supérieur à la fraude aux prestations sociales. Ainsi, le non-recours pour le revenu de solidarité active (RSA) est de 36 soit plus de 3,6 milliards d'euros ; le non-recours pour la couverture maladie universelle est de 34 % ; enfin, le non-recours pour l'aide à la complémentaire santé Dans le Pas-de-Calais, des familles survivent sous les radars et renoncent à leurs droits, car elles refusent d'être stigmatisées et considérées Nos concitoyens renoncent à leurs droits par méconnaissance et parce qu'ils sont montrés du doigt. Cette proposition de loi stigmatise les plus pauvres au lieu de s'attaquer aux riches et aux puissants, véritables fraudeurs professionnels.

matière depuis de longues années, nous propose aujourd'hui de légiférer afin d'appliquer des mesures urgentes de lutte contre la fraude sociale. Le champ de la fraude est si vaste, si complexe, si évolutif qu'il est délicat de choisir les outils les plus efficaces, les plus pertinents, les plus opérationnels. C'est ainsi que le texte initial, volontairement limité au champ de la fraude sociale, a été recentré par la commission, sur proposition du rapporteur, sur quelques sujets cibles, qui permettront au Parlement d'émettre un signal fort. En effet, la fraude en général est, par essence, insupportable et inadmissible. Nous ne pouvons la tolérer. Lutter contre les fraudes, c'est défendre notre contrat social. S'il subsiste des incertitudes sur le volume financier réel de la fraude, une chose est certaine, c'est que les sommes non collectées ou distribuées à tort ne pourront plus être affectées, directement ou indirectement, à la politique sociale. Le système français de sécurité sociale se caractérise par sa diversité et son extrême complexité dans la délivrance des prestations sociales. Il fonctionne par traitements de masses et dématérialisation de l'information. Il doit désormais faire face à des populations qui ne sont plus attachées strictement à un territoire. Tout cela ouvre, hélas, une large porte à des réseaux de fraude, aux systèmes très organisés. Les fraudes sociales touchent à l'identité, à la composition familiale, aux liens de parenté, au décès, à la nationalité, à la résidence, à l'état de santé, au niveau de revenus, etc. Elles se caractérisent par l'obtention indue de droits à l'assurance maladie, à l'aide médicale de l'État, à des prescriptions, à des cumuls de prestations, etc. Alors que les systèmes de fraude évoluent avec une agilité déconcertante, la réglementation et la loi doivent, avec la même agilité et la même rapidité, produire les parades adaptées. « La police doit aller aussi vite que les voleurs », nous disait il y a peu Gérald Darmanin. Eh bien, il doit en Aussi, au-delà de ce texte examiné en ce 11 mars 2021, mes chers collègues, je crois sincèrement que nous devons nous préparer à remettre sans cesse sur le métier cet ouvrage et nous retrouver aussi souvent qu'il le faudra pour voter de nouvelles mesures urgentes de lutte contre la fraude sociale. Nous le ferons, parce que frauder, c'est voler.

c'est qu'est bien fini le temps des « fraudo-sceptiques », le temps où le sujet était pudiquement glissé sous le tapis. Il faut désormais prendre le problème à bras-le-corps, s'en saisir et ne plus jamais détourner le regard. Cela passe certainement par des moyens en matériel et en personnel indispensables.

d'action volontariste. Dans la mesure où tout document peut être falsifié et sachant que la fraude documentaire est la mère de toutes les fraudes, j'insiste sur l'utilité absolue de disposer de documents d'identification en couleur et de qualité correcte.

viens aux retraites versées à étranger. Pour mettre fin à des dérives connues et scandaleuses, il faut sécuriser les données de certificats de vie en utilisant des données biométriques et en conventionnant avec les organismes de retraite d'États étrangers.

qui, pour être indemnisés de leurs prestations dans les centres de vaccination covid, doivent produire un dossier très complet, avec extrait Kbis, casier judiciaire et déclaration de situation matrimoniale -, alors que, parallèlement et grâce à tout cela,

doit être menée de front. Vous avez compris, et Mme Goulet l'a rappelé dans son propos liminaire, que le volume de recettes que nous pouvons récupérer par la lutte contre la fraude

puissent les faire valoir. C'est d'ailleurs parce que nous arriverons à faire payer ceux qui peuvent payer leurs cotisations que nous pourrons encore mieux financer l'accès aux droits de ceux qui en ont besoin et qui y ont légitimement accès.

outre le fait que je n'en partage pas l'orientation générale. D'une part, vous avez indiqué que la France avait perdu 700 000 emplois en 2020. C'est totalement faux : nous avons perdu 360 000 emplois, ce qui est évidemment beaucoup trop. Nous craignions d'en perdre 900 000. Quand on traverse une crise économique, il ne faut pas dramatiser ou ajouter du pessimisme à la situation que l'on connaît. part, l'Insee a rendu publiques ses estimations sur l'année 2020 et sur le quatrième trimestre de cette même année. Il se trouve que, de manière globale, c'est-à-dire en moyenne, et je n'ignore rien des disparités de situation, le pouvoir d'achat des ménages français a augmenté de 0,6 % en 2020.

à écouter tous les orateurs, j'ai bien compris l'intérêt que chacun portait à la question des documents d'identité en couleur pour éviter la fraude documentaire. C'est un sujet sur lequel nous travaillons et pourrons avancer, y compris de manière réglementaire, pour faire en sorte de mieux prévenir et d'éviter la falsification des documents. Je précise par ailleurs que la falsification des documents est souvent l'un des piliers de la fraude organisée. Bien souvent,

Le non-recours aux prestations est un fléau bien plus répandu, notamment en matière d'accès aux soins, que la fraude sociale et l'intérêt pour ce sujet, en particulier de la majorité sénatoriale, est bien moins important et aucunement à la hauteur du phénomène. Pourtant la question du non-recours nous interroge sur l'effectivité et la pertinence de nos politiques publiques de protection sociale, ainsi que sur la place accordée à l'usager dans l'action publique. Elle est outre un enjeu fondamental de leur évaluation. C'est pourquoi nous sommes en droit d'attendre de la commission des affaires sociales du Sénat, qui a consacré, sur l'initiative de la majorité sénatoriale, plusieurs rapports d'information à la fraude sociale, qu'elle montre la même ténacité à prendre à bras-le-corps

aux amendements identiques de suppression présenter l'amendement n° 11. L'article 4 de cette proposition de loi autorise l'accès aux données des plateformes en ligne pour contrôler les assurés sociaux au détriment, de notre point de vue, des libertés individuelles et du respect de la vie privée. Tout d'abord, permettez-moi de rappeler que, concernant l'usage des fichiers et de leur croisement pour renforcer les contrôles, la CNIL autorise « l'automatisation des outils, mais le croisement des données et les requêtes ne doivent pas prendre la place de l'intervention humaine dans le schéma de décision ».

que « le développement des contrôles depuis une dizaine d'années et les pouvoirs nouveaux conférés aux régimes de protection sociale et à Pôle emploi ne sont pas sans soulever un certain nombre de questions de questions ». En effet, le renforcement des contrôles entraîne un accroissement du nombre de réclamations, car « la politique mise en oeuvre en la matière, marquée par certains excès et quelques dérives, [est] la source de nombreuses atteintes aux droits des usagers des services publics ». Enfin, le recours croissant Enfin, le recours croissant au, qui établit d'éventuelles corrélations signifiantes et utilisables entre les données, peut lui aussi poser des problèmes, la définition des profils ou des situations à risques n'étant évidemment pas neutre. La sécurité sociale dispose déjà des outils pour lutter contre la fraude, mais, on le voit, tout n'est pas réglé. Elle manque de moyens humains : ce sont eux qu'il faut renforcer. La proposition de loi visant à lutter contre la fraude aux prestations sociales ne cherche donc pas à améliorer les contrôles, de notre point de vue, mais plutôt à renforcer les conditions d'accès aux prestations sociales, ainsi que la mise en place d'une cybersurveillance. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

qu'on puisse proposer à l'encontre des personnes bénéficiaires des prestations sociales des mesures de collecte et d'exploitation de leurs contenus librement accessibles sur internet, notamment sur les réseaux sociaux, et pas seulement du fait de la complexité de la mise en oeuvre d'une telle mesure, mais parce que l'État de droit garantit la protection des données à caractère personnel. Pour les écologistes, il s'agit d'un pas de plus vers la surveillance des personnes sur internet, en collectant des contenus relatifs à la vie privée. Rappelons que la CNIL s'était déjà montrée critique lorsque le Gouvernement avait suggéré un dispositif similaire ouvrant cette possibilité à l'administration fiscale et douanière loi de finances de 2019, en s'interrogeant sur son opportunité au regard des garanties fondamentales d'exercice des libertés publiques. Aussi, nous devrions nous soucier de la conformité de cet article au RGPD. Je rappelle également que les publics ciblés par les prestations sociales font déjà l'objet de différents contrôles. Pour le RSA, par exemple, des départements déploient leurs propres contrôles, en plus de ceux de la CAF et de Pôle emploi. Ces trois instances sont déjà dotées de moyens de contrôle, et il convient de rappeler que leur rôle premier est d'accompagner, de permettre l'accès aux droits des personnes en difficulté, ce qui suppose au préalable d'installer une relation une relation de confiance. Les moyens de surveillance généralisée renversent ce positionnement, et ce n'est pas acceptable. Trop souvent, l'obsession de la chasse aux fraudeurs fait vivre aux personnes concernées des calvaires administratifs aux conséquences quelquefois graves, quand elle n'a pas pour principal effet le renoncement aux droits. Nous n'avons donc pas besoin d'un dispositif de surveillance supplémentaire qui se montrerait encore plus intrusif, au mépris des libertés individuelles, du respect des données et de la vie privée des personnes en situation de précarité. Pour un cas, combien de personnes, sur les 7 millions de personnes concernées par un minima social, seront ainsi malmenées ? Nous proposons, par cet amendement, la suppression de cet article, et pas seulement de voter contre.

de contrôle pour lutter contre la fraude au RSA. Il ne nous paraît pas utile d'aller au-delà. Ces bases nous paraissent suffisantes pour permettre les échanges utiles dans le cadre des Codaf en particulier, puisque les conseils départementaux sont invités au cas par cas et en fonction de l'ordre du jour. Nous ne sommes donc pas favorables à cette extension des prérogatives des agents habilités par les conseils

Mme Cathy Apourceau-Poly. L'article 8 renforce drastiquement les conditions d'accès à l'APL, en subordonnant le versement de cette aide à la transmission d'informations sur le logement. telle mesure complexifie inutilement la procédure aux dépens des droits des familles les plus précaires. Je rappelle que, en 2019, l'omission constituait 70 % des fraudes détectées, tandis que la production et l'usage de faux documents représentaient seulement 12,5 des fraudes qualifiées. Alors que le Gouvernement a institué pour les entreprises un droit à l'erreur, vous proposez d'inverser la charge de la preuve pour les plus pauvres, soumis à la suspicion permanente de la tentative de fraude. La réalité, c'est que, à force de renforcer les contrôles pour prétendument plus de justice, vous découragez les honnêtes citoyens qui pourraient bénéficier des aides sociales. Aujourd'hui, le non-recours est renforcé par les multiples démarches administratives imposées prétendument pour vérifier l'absence de fraude. C'est le constat du rapport du Secours catholique pour l'année 2018, qui indiquait une baisse de l'accès aux allocations familiales de 5 83 % de ces familles percevaient les allocations familiales en 2010 et seulement 78 % en 2017. En limitant la lutte contre la fraude aux prestations sociales des assurés sociaux, le texte stigmatise les plus précaires et refuse de s'attaquer à la fraude des entreprises, dont le montant est évalué par la Cour des comptes à 25 milliards d'euros, soit 25 fois plus que le montant total de la fraude aux prestations et 250 fois celle de la « fraude documentaire ». Tel est le sens de cet amendement de suppression. Quel

de suppression de l'article 8, parce qu'il nous paraît intéressant d'avoir des précisions sur le logement auquel l'aide se rapporte.

l'avis du Gouvernement ? L'objectif visé par cet article est de sécuriser le versement des aides au logement, ce qui paraît légitime et souhaitable. Toutefois, subordonner le versement de l'APL à la transmission aux CAF des principales caractéristiques du logement auquel l'aide se rapporte, susceptible d'affecter sa valeur locative, n'a pas réellement d'intérêt en termes de contrôle. En effet, cette valeur locative n'est pas prise en compte dans le calcul de l'aide au logement et ne peut donc servir à détecter une fraude. Le Gouvernement ne peut retenir cette mesure en l'état. Il est donc favorable à cet amendement de suppression. Je mets aux voix

: La parole est à Mme Corinne Imbert. Cet amendement vise à prévoir un changement de procédure d'attribution du RSA à compter du 1 janvier 2023. Il ne reviendrait plus au demandeur de fournir les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande, mais à l'administration ou à l'organisme

partage tout à fait l'intention exprimée par notre collègue. Elle s'interroge cependant sur les possibilités qui existent déjà pour les services en matière d'information pour instruire les demandes au sein des CAF.

les données nécessaires à l'examen des demandes auprès des autres administrations sans qu'il soit utile de compléter le code de l'action sociale et des familles en ce sens. Par ailleurs, des travaux sont engagés en ce moment même pour que les CAF et les caisses de la MSA puissent récupérer les informations sur les ressources des demandeurs auprès des différents opérateurs impliqués. Cette réforme est rendue possible par la disponibilité des données issues des déclarations des employeurs et des organismes qui versent des prestations sociales. La récupération automatique des ressources des bénéficiaires se fera par le biais du dispositif de ressources mensuelles créé par l'article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Cela permettra de simplifier les démarches des déclarants, de stabiliser les droits versés en limitant les indus et les rappels, de faciliter la gestion pour les caisses et de favoriser le juste recours à la prestation. Cet amendement apparaît donc satisfait en droit et le sera très prochainement en pratique par une récupération désormais automatique de certaines données. Le Gouvernement estime donc qu'il est satisfait : il en demande le retrait ; à défaut, l'avis sera défavorable. Madame Imbert,

en 2021 ! C'est une application du « dites-le-nous une fois » : on remplace le déclaratif par un échange et une inversion de

pensionnés résidant à l'étranger ou dans certains territoires ultramarins. À l'occasion de cette codification, nous avons également ouvert la possibilité de recourir à la biométrie pour assurer le contrôle de l'existence.

Le rapporteur avait consulté sur ce sujet la CNAV, l'Agirc-Arrco, le GIP Union Retraite pour mieux comprendre la répartition des rôles et le fonctionnement de ce contrôle de l'existence au sein des caisses. La rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ne me semble pas devoir être modifiée aujourd'hui, d'autant que, comme je l'ai déjà évoqué, l'intention de l'auteur de la proposition de loi est tout à fait satisfaite par les dispositions qui sont issues de cette loi. Les organismes concluent déjà des conventions avec leurs homologues à l'étranger, permettant notamment des échanges automatisés d'état civil. La présente rédaction ne contraint pas davantage les procédures ni n'ouvre de faculté nouvelle. Nous vous invitons donc

En fait, je souhaitais intervenir sur l'article 9 relatif aux échanges d'informations entre organismes européens de sécurité sociale. La commission des affaires sociales a jugé bon de le supprimer, considérant qu'un règlement européen portant coopération des systèmes de sécurité sociale les prévoyait déjà. Les prévoir dans la législation française ne serait donc plus nécessaire, selon la commission ... À titre personnel, je ne suis pas sûr que cette coopération entre organismes européens de sécurité sociale soit efficace à 100 %. J'aimerais J'aimerais redire ici qu'en zone frontalière la fraude sociale est une réalité et qu'il convient de lutter plus fermement contre son développement. Or cette fraude est rendue possible, voire facilitée par l'absence ou l'insuffisance d'échanges de données entre les pays et les organismes sociaux, même si de nombreux progrès ont été réalisés au fil des années depuis ce règlement. Une meilleure coopération entre administrations des pays concernés est essentielle, en attendant peut-être à terme une harmonisation complète au niveau européen de nos systèmes de protection. La commission des affaires européennes poursuit un travail important en ce sens, et j'ai moi-même eu l'occasion, en janvier 2020, de déposer une proposition de résolution européenne visant à lutter contre la fraude aux prestations sociales et mettant l'accent sur l'urgence de renforcer la coopération entre les États. Celle-ci a été adoptée par notre commission des affaires européennes en février 2020, ce qui montre que tout n'est pas parfait en la matière, c'est le moins qu'on puisse dire. Je voudrais également dire un mot de la suppression, par la commission, de l'article 11, qui proposait à l'origine qu'un décret établisse une liste de pays dont l'état civil serait présumé non fiable. Si, comme l'a dit la commission, le dispositif proposé risquait de poser des problèmes diplomatiques ou politiques sans vraiment résoudre le problème posé, je voudrais, en qualité de président du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest, confirmer ici les faiblesses administratives que connaissent certains pays de la zone en matière d'état civil et, dès lors, confirmer les risques importants de fraude à l'identité que cette situation génère. Il est donc indispensable que la lutte contre cette fraude passe par un encouragement des États concernés à se doter au plus vite des instruments permettant la tenue d'un état civil rigoureux et fiable. Mes chers collègues, socialement, la fraude n'est plus acceptable, surtout dans le contexte difficile que nous connaissons. En tant que parlementaires, nous devons nous atteler à éliminer toutes ces formes de fraudes, qui réduisent par leur existence même nos capacités budgétaires. Je tiens donc à féliciter et à remercier Nathalie Goulet et ses collègues de leur initiative.

de moyens pour lutter contre la fraude au paiement des cotisations sociales. Les plans d'économies, année après année, ont dépecé les services de l'encaissement des cotisations sociales. il faut un engagement politique, financier et humain pour lutter contre la fraude aux cotisations patronales, estimée à 25 milliards d'euros par la Cour des comptes. Par cohérence avec l'objet de la proposition de loi, qui mentionne la fraude sociale, nous demandons que le Gouvernement réalise une évaluation récente sur le montant de la fraude patronale aux cotisations sociales et, surtout, formule des recommandations pour lutter contre ce type de fraude. L'avis défavorable de la commission des affaires sociales démontrera bien que vous refusez de vous attaquer au coeur du problème et préférez pointer du doigt les plus pauvres de ce pays. Quel commission ? Je conteste tout à fait les conclusions de Mme Apourceau-Poly : nous ne stigmatisons pas plus les pauvres que les entreprises dans cette affaire. Un tel rapport ne nous semble pas présenter d'utilité particulière.

régulièrement. Le rapport sur les fraudes transfrontalières que nous venons de voter à l'article 12 peut d'ailleurs mettre en lumière certaines de ces techniques et les moyens d'y remédier. Pour l'heure, la commission

de disposer de plus d'informations pour mieux évaluer la réalité de la fraude sociale sous toutes ses formes. Le montant du manque à gagner résultant pour la sécurité sociale des cotisations éludées par les employeurs fait d'ailleurs, vous le savez,

Évidemment, de nouvelles estimations de la fraude seront réalisées par l'Acoss et par la CCMSA dans le cadre du plan Fraude lancé en janvier. Cet effort renouvelé pour disposer de chiffres fiables sur la fraude sociale sous toutes ses formes

L'article 14 rend obligatoire la création d'un compte bancaire en France pour obtenir le versement des prestations sociales. Cette contrainte administrative inutile est stigmatisante pour les personnes étrangères, qui devront payer les frais d'ouverture et de gestion d'un compte bancaire pour bénéficier de l'aide sociale. Cette disposition est d'autant plus inacceptable que, s'agissant des entreprises, le Gouvernement ne demande pas, pour verser l'aide du fonds de solidarité, de disposer d'un compte bancaire en France. Le fonds de solidarité pour prévenir la cessation d'activité des entreprises touchées par les conséquences économiques du covid-19 prévoit, je cite : « Tous les comptes, domiciliés dans un établissement bancaire en France ou à l'étranger, sont acceptés par le formulaire. L'article 14 va donc créer une inégalité de situation entre les entreprises et les bénéficiaires des aides sociales, puisque les premiers n'ont pas d'obligation de disposer d'un compte bancaire financier en France pour toucher l'aide financière de l'État. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article. Quel

Au demeurant, le dispositif serait encore plus efficace si l'obligation de versement se limitait aux comptes français, mais cela contreviendrait au droit communautaire, comme le Gouvernement nous le confirmera sans doute. La commission a souhaité conserver cet article. Elle a donc émis un avis défavorable à sa suppression par le groupe CRCE.

permettrait de contrôler l'identité des titulaires de comptes bancaires. Le droit européen, qui interdit de traiter différemment les établissements bancaires établis dans l'Union, et l'absence d'outil de type Ficoba à l'échelon communautaire vident en pratique la mesure proposée à l'article

cet outil de la flagrance permet aux agents des impôts de dresser un procès-verbal qui emporte des effets comme des mesures conservatoires en cas de constatation de faits frauduleux. Rapide et efficace, la flagrance a fait ses preuves dans la lutte contre la fraude fiscale. Cet amendement tend donc à créer la flagrance sociale, un outil à disposition des inspecteurs de recouvrement, afin de percevoir les prestations sociales obtenues frauduleusement.

de montrer que l'assuré a sciemment minoré le montant de ses revenus, par exemple pour bénéficier d'une prestation sous conditions de ressources. D'autre part, le recouvrement des indus frauduleux se heurte très souvent bien plus à l'insolvabilité de l'assuré qu'à la difficulté de saisir des biens, comme c'est le cas pour une entreprise fraudant aux cotisations et organisant son insolvabilité. La procédure ne semble donc pas adaptée aux fraudes sociales

confèrent déjà à des agents chargés du contrôle agréés et assermentés le soin de procéder à toute vérification ou enquête administrative concernant l'attribution des prestations ou le respect des conditions de résidence, de ressources, etc. Cela implique la possibilité de convoquer physiquement la personne objet du contrôle. En d'autres termes, les

présenter l'amendement n° 14. L'article 18 habilite les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et de l'inspection du travail à mener des enquêtes judiciaires. Il n'est pas acceptable de transférer la mission des services d'enquête judiciaire

Étendre encore l'habilitation aux fraudes des prestations sociales revient à faire supporter une partie du coût des enquêtes aux organismes de protection sociale. Surtout, cela désengage en fait l'État de ses responsabilités. En matière fiscale, la création de la procédure judiciaire d'enquête fiscale s'est accompagnée de celle de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, composée d'officiers de police judiciaire et d'agents des services fiscaux. L'article 18 prévoit de confier aux agents de contrôle de la sécurité sociale et de l'inspection du travail une mission qui nécessiterait la création d'un corps distinct avec des personnels formés spécifiquement à la procédure pénale.

Le discours récurrent sur la fraude sociale tend en effet à faire croire que notre système serait en lui-même « fraudogène » et à alimenter la suspicion vis-à-vis de ceux qui en bénéficient légitimement. Or nous bénéficions tous à un moment de notre vie, à un degré ou à un autre, de prestations sociales. Si la lutte contre la fraude intentionnelle est légitime, elle se doit d'être juste. D'abord, elle doit nécessairement s'accompagner du même volontarisme en matière d'accès aux droits et de lutte contre le non-recours aux prestations sociales. viser tous les types de fraudes, en premier lieu la fraude fiscale, qui est bien supérieure en termes de montants à la fraude sociale. Cessons de faire croire que la fraude aux prestations est plus importante que la fraude aux cotisations. C'est l'inverse qui est vrai : les entreprises et les professionnels fraudent plus que les particuliers. En conséquence, n'allons pas au plus facile en visant prioritairement les particuliers. Sortons de l'amalgame que le vocable « fraude sociale » suggère entre les situations individuelles qui relèvent de la non-intentionnalité et qui sont essentiellement dues à la complexité administrative du système de protection sociale et les fraudes intentionnelles, organisées, au premier rang desquelles celles des réseaux « professionnels », qui relèvent, elles, de la délinquance.

la fraude patronale était estimée entre 6,8 milliards et 8,4 milliards d'euros, soit huit fois plus que la fraude aux prestations sociales.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à titre liminaire, je voudrais remercier l'ensemble des membres de la commission mixte paritaire, qui s'est réunie le 2 mars dernier.

sans consultation préalable de l'Assemblée nationale, ni des forces politiques, ni encore du Conseil d'État. Le procédé a d'ailleurs fortement ému non seulement les sénateurs, mais également les députés, considérant qu'il s'agissait là d'une question de respect du Parlement et, plus largement, de nos institutions. Dans ces conditions- tout le monde en conviendra -, il était singulièrement difficile d'aborder une telle problématique.

la réflexion doit être totalement déconnectée de tout contexte électoral, en particulier de l'élection clé de voûte de nos institutions.

il semble indispensable de prendre beaucoup de recul pour mesurer dans un climat serein et apaisé toutes les conséquences d'idées qui peuvent paraître novatrices, modernes,

l'accord des deux chambres sur un texte commun nous a paru tout à fait possible. D'ailleurs, certains apports non négligeables du Sénat n'ont soulevé aucune difficulté. J'en mentionnerai cinq. Le premier de la campagne électorale aux personnes en situation de handicap. C'est vraiment une avancée majeure. Certes, nous restons au stade de l'incitation pour l'ensemble des candidats, tout en nous appuyant sur l'expertise du Conseil national consultatif des personnes handicapées. En effet, la multitude des supports de propagande et la diversité des handicaps ne nous ont pas permis d'aller plus loin.

Le quatrième est le caractère expérimental de la dématérialisation des comptes de campagne et des reçus-dons, qui permettra d'évaluer le dispositif avant toute généralisation éventuelle.

Implicitement, cela permettra de sécuriser la période dite « intermédiaire » tout en laissant un laps de temps suffisant au Conseil constitutionnel pour contrôler les parrainages.

Celle-ci était fixée à un an, contre six mois pour les autres élections.

proposition avait un objectif clair : éviter tout chevauchement avec les élections régionales et départementales qui auront lieu au mois de juin prochain.

à la députation. Incontestablement, nous ne sommes pas dans la même chronologie. Le délai d'un an avait été maintenu pour l'élection présidentielle afin d'englober les primaires. Or aucun parti n'a prévu l'organisation de primaires d'ici au 1 juillet prochain. Le délai de neuf mois, qui correspond d'ailleurs à l'idée initiale du Gouvernement, nous semble donc le plus adapté pour la prochaine

Le texte qu'il vous est proposé de voter cet après-midi et auquel le Gouvernement donnera un avis favorable nous invite à l'inverse à en terminer avec le dérogatoire et à nous projeter résolument vers l'avenir,

qui a présidé à vos débats lors de l'examen de ce projet de loi organique. Ces travaux ont été empreints d'une grande gravité, cette gravité qui sied lorsque nous touchons collectivement à la matière électorale, à la fois technique et pourtant ô combien structurante pour notre fonctionnement collectif. Comme le disait le juriste allemand von Jhering, la procédure est soeur jumelle de la liberté. En droit électoral, les règles déterminées par le législateur sont bien les garantes d'un scrutin chaque fois sincère, transparent et démocratique, et, comme chaque année qui précède le scrutin présidentiel, la loi organique qui en adapte les règles ressort de l'examen parlementaire non pas dénaturée, mais enrichie et consolidée. À cet égard, vous avez À cet égard, vous avez finalement décidé de limiter à neuf mois la durée de la campagne présidentielle- vous le savez, ce n'était pas la volonté originelle du Gouvernement. Gouvernement. Votre souci de sécuriser la computation des comptes de campagne pour cette période 2021-2022 un peu exceptionnelle, où les scrutins régionaux, départementaux et présidentiels se suivent, si bien que les campagnes

de tous les majeurs sous tutelle et qui prévoit la production par les candidats de professions de foi en langage dit facile à lire et à comprendre pour l'élection présidentielle. C'est l'objet de l'article 1 , adopté par votre assemblée, qui rehausse notre vigilance collective sur ces sujets, et c'est heureux. La participation la plus large possible, c'est aussi plusieurs mesures ambitieuses qui figurent dans ce projet de loi organique. Je pense notamment à la déterritorialisation du vote par procuration, qui sera appliquée pour la première fois dans notre pays lors de ce scrutin, avant d'être généralisée, comme prévu, à l'ensemble des élections. S'appuyant sur le répertoire électoral unique pleinement opérationnel à compter du 1 janvier 2022, elle permettra de recourir beaucoup plus facilement au vote par procuration sans rien enlever à l'impératif de sécurité. Je rappelle à ce sujet que nos nos concitoyens pourront également profiter du dispositif déployé en ce moment par le ministère de l'intérieur dénommé e-procuration, qui dématérialise l'essentiel de la procédure de demande et de transmission en mairie de ces procurations.

Qu'apporte-t-il ? Le rapporteur l'a rappelé : quelques avancées en matière de date de publication du décret de convocation des électeurs, de procédure de parrainage des candidats

Nous avons également obtenu que la diffusion de certains sondages d'opinion soit accompagnée des marges d'erreur. Le seul vrai problème de la discussion de ce texte a été

Le vrai souci de cette proposition, c'est qu'elle a délégitimé le vote anticipé, en passant par une modalité improbable d'utilisation des machines à voter, alors même que le moratoire sur celles-ci n'est toujours pas levé et qu'un rapport devait être rendu sur le sujet. le sujet. Si ce toilettage technique était nécessaire, nous sommes à nouveau restés en deçà de ce qui aurait été utile. En démocratie, la règle est simple : le pouvoir politique s'exerce selon des règles et des procédures préalablement fixées et établies.

Si, pour reprendre l'expression de Benjamin Barber, il faut avoir une conception « forte » de la démocratie, celle-ci passe nécessairement par l'évolution du droit électoral. Ces évolutions auraient été emblématiques pour le scrutin qui, à tort ou à raison, reste le premier rendez-vous démocratique en France.

Philippe Ardant notait que « toute l'histoire du régime représentatif suggère une évolution linéaire vers une plus grande démocratie par un élargissement constant du nombre et des catégories d'individus appelés à participer au rituel du choix des représentants ». Pourtant, rien n'est plus faux que cette impression.

Le droit électoral est un enjeu démocratique comme politique. Il est un enjeu politique, quand on tend de fait, comme dans le sud des États-Unis, à réduire la capacité d'expression de certains groupes, essentiellement les minorités, en les privant du droit de vote par tous les moyens dans le but d'empêcher d'empêcher le changement politique. Il est un enjeu démocratique, quand on constate l'autoexclusion, qu'elle soit volontaire ou pas, d'une partie de l'électorat, que l'on parle des non-inscrits,

que l'on parle de tous ceux qui ne s'estiment pas compétents pour donner leur avis, de ce « cens caché » qui peut exister au sein de notre démocratie. Oui, pour détourner la parole de Pierre Bourdieu, le droit électoral, comme la sociologie, est un sport de combat, parce qu'aucune voix ne devrait peser plus qu'une autre, alors que c'est de fait le cas, notamment au travers des règles de financement électoral qui existent dans notre pays. Il n'est pas indifférent que la mesure d'adaptation du droit électoral privilégiée

Bien entendu, certains me diront que des dispositions techniques ne suffisent pas à répondre aux défis démocratiques de la démobilisation électorale. J'en conviendrai aisément avec eux. Mais considérer que de tels aménagements n'ont aucun effet sur la participation est tout aussi faux. Si la participation baisse avec le grand âge, alors le vote par correspondance peut être une réponse. Il ne s'agit pas de remettre en cause le rite républicain du vote, qui demeure intégrateur, mais de le revigorer. Las, par paresse, la majorité sénatoriale a refusé l'ensemble des évolutions que nous avions proposées, en s'abritant derrière la timidité du rapport d'information sur le vote à distance. Comme ce n'est pas le bon moment, ce n'est jamais le moment ! Nous aurions pu être des aiguillons ; nous serons des techniciens craintifs. Nous voterons ce texte, parce qu'il contient de petites avancées utiles, mais nous le ferons sans le moindre enthousiasme. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je me réjouis que la commission mixte paritaire soit parvenue à une rédaction commune de l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République. particulièrement heureux qu'elle ait retenu l'ensemble des apports du Sénat. Je pense notamment aux dispositions visant à améliorer les règles de propagande électorale : renforcement de l'accessibilité de la propagande aux personnes en situation de handicap ; obligation pour les instituts de sondage de publier leurs marges d'erreur lors de toute publication ou diffusion d'un sondage relatif à l'élection présidentielle ; fixation d'une date plus précoce pour la publication de la liste des candidats, ce qui permet de sécuriser la période intermédiaire, pendant laquelle les médias doivent donner la parole de manière équitable à l'ensemble des candidats et dans des conditions de programmation comparables. Je pense également aux mesures qui tendent à adapter les règles de financement de la campagne : faire débuter la période de financement de l'élection présidentielle au 1 juillet 2021 pour une durée d'environ neuf mois ; augmenter l'avance versée à l'ensemble des candidats pour faciliter le financement des campagnes et tenir compte de l'inflation ; conférer un caractère expérimental à la dématérialisation des comptes de campagne de l'élection présidentielle et des reçus-dons reçus-dons ; publier les comptes de campagne de l'élection présidentielle en. Je pense enfin aux dispositions relatives à la sécurisation de l'organisation de l'élection présidentielle : convocation des électeurs par décret simple ; actualisation de la liste des parrains pouvant présenter un candidat ; amélioration du fonctionnement des commissions de contrôle qui veillent à la régularité des listes électorales consulaires des Français de l'étranger.

Notre assemblée s'y est fermement opposée, et je m'en félicite. Il s'agissait d'une question de respect du Parlement et, par là même, de nos institutions. Sur la forme, l'amendement du Gouvernement a été déposé devant la seconde chambre saisie, sans consultation préalable des forces politiques ou du Conseil d'État et sans que l'Assemblée nationale ait été appelée à se prononcer.

Comment garantir la sécurité des machines à voter ? Où auraient-elles été disposées ? Sous quelle responsabilité auraient-elles été placées ? Si nous ne refusons pas de réfléchir à des évolutions de notre droit électoral, une telle réflexion doit se faire de manière apaisée, à bonne distance des échéances électorales. Madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi organique qui nous est soumis a été conçu comme un texte de réglage comprenant divers ajustements techniques. Il s'inscrit dans la continuité des textes de toilettage adoptés avant chaque élection présidentielle depuis 1988 pour mettre en conformité les mesures d'organisation de l'élection présidentielle avec les évolutions du code électoral. Aussi, le groupe Les Indépendants le votera. La parole

il a assez fait parler de lui- trop, vraisemblablement ! Je vais commencer par saluer les quelques avancées techniques, qui sont essentiellement dues à la sagesse des parlementaires, lesquels ont su s'accorder sur un texte qui avait été travaillé de manière assez équilibrée par notre commission et notre assemblée. Comme l'a déjà fait remarquer notre rapporteur, le texte reprend les avancées prévues par nos travaux sénatoriaux. Toutefois, je continue de regretter l'abandon de la transmission électronique des parrainages, pourtant prévue depuis plusieurs années et repoussée à l'élection

ce texte prévoit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mette en oeuvre un téléservice permettant l'édition et la délivrance de reçus pour chaque don versé à un candidat et un autre pour recevoir de manière dématérialisée les comptes de campagne. évidemment que cette simplification numérique bénéficie des mêmes critères de sécurité qui justifient le non-recours à la dématérialisation des parrainages J'en profite pour souligner l'importance fondamentale d'un sujet peu souvent mis en avant : le vote des détenus. Je l'ai déjà dit, mais je souhaite le répéter : la prison est certes le lieu d'exécution de la peine, mais elle est aussi le lieu qui doit permettre la réinsertion du délinquant. Comment envisager une réinsertion, alors que ces personnes sont exclues de fait, et non en droit, de la participation à la vie citoyenne que constitue le moment fort de notre vie démocratique, l'élection présidentielle ? Malgré le succès relatif de l'établissement de bureaux de vote lors des élections européennes, il a été choisi de ne pas renouveler l'expérience pour se concentrer sur le vote par correspondance. Il est dès lors très important que l'administration pénitentiaire prenne part activement à l'information des détenus sur leur droit à être inscrits sur une liste électorale, mais aussi sur les démarches à effectuer et sur les modalités du vote par correspondance. Le texte a aussi gardé les modifications sur le vote par procuration, considéré comme une modalité du vote ne nécessitant plus d'être justifiée et devant s'appliquer à tous, y compris aux Français de l'étranger.

le fait que les apports sénatoriaux sur les conditions de publication des sondages aient été conservés. Certes, d'un point de vue personnel, mes réticences sur les dates possibles de ces publications sont bien plus grandes. Il n'en reste pas moins que notre texte permet d'apporter une explication de ces chiffres, de montrer les limites des méthodes statistiques sur les intentions de vote et d'accompagner ces publications des marges d'erreur calculées, voire de réglementation plus drastique sur les périodes tolérées de réalisation et de diffusion.

Notre système est à bout de souffle, notre démocratie fragilisée, pas seulement en raison des mesures restrictives prises au nom de la lutte contre la pandémie. Il est donc plus que temps de réfléchir sur notre République et sur les dangers de l'hyperprésidentialisation. La légitimité issue des citoyens ne devrait pas pouvoir être détachée de la responsabilité envers eux- les deux sont liées. Le Président, en gouvernant seul, hors du cadre régulier prévu par notre démocratie, se permet en quelque sorte d'échapper aux électeurs. Les tentatives maladroites d'établissement de nouveaux contours pour l'élection au coeur de notre système, à l'image de l'exercice singulier, sous bien des aspects, de la présidence de la République actuelle, ne sont pas de notre goût. C'est pourquoi le groupe GEST ne pourra pas voter ce texte : il abstiendra.

Bien que notre pays traverse encore des difficultés liées au contexte sanitaire qui nous ont poussés à adapter nos différents rendez-vous démocratiques, récemment les élections régionales et départementales, ce projet de loi organique en finit avec le cadre dérogatoire et nous projette vers un retour à la normale. Le groupe RDPI se félicite que la réunion de la commission mixte paritaire ait pu déboucher sur un accord concernant ce texte de réglage et de coordination pour le prochain scrutin présidentiel de 2022. Il nous revient aujourd'hui d'en valider les conclusions et de souligner la qualité du travail réalisé par les deux chambres, ainsi que les différents apports et innovations qui bénéficieront aux électeurs et aux candidats pour garantir un scrutin toujours plus sincère, transparent et démocratique. Comme ont pu le rappeler certains collègues, ce texte vise essentiellement à actualiser des dispositions de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. D'une part, il apporte des précisions et des innovations pour les électeurs afin de créer les conditions de participation la plus large possible à ce scrutin. Je pense notamment à la publication du décret de convocation des électeurs et au vote par procuration des personnes détenues, qui a été expérimenté dans le cadre des élections européennes de 2019. Conformément à la loi Engagement et proximité, le texte prévoit la déterritorialisation des procurations. Il procède aussi à l'adaptation de dispositions relatives aux listes électorales consulaires et au vote des Français de l'étranger. D'autre part, le texte actualise la liste des parrains pouvant présenter un candidat à l'élection présidentielle, en tenant compte des dernières réformes territoriales et en y ajoutant les 152 présidents des conseils consulaires des Français de l'étranger. Le texte que nous votons adapte aussi les règles de financement pour éviter tout chevauchement avec les comptes de campagne des élections régionales et départementales de juin 2021, pour expérimenter la dématérialisation des comptes de campagne de l'élection présidentielle et des reçus-dons et, enfin, pour publier les comptes de campagne de l'élection présidentielle en. À cela À cela s'ajoute une autre avancée majeure concernant la propagande électorale. Les candidats auront de nouvelles obligations en matière d'accessibilité de leur campagne : ils devront tenir compte des différentes formes de handicap et de la diversité des supports de communication, comme suggéré par notre collègue Philippe Mouiller. Pour finir, permettez-moi de revenir sur le vote par anticipation proposé par le Gouvernement. Certes, la méthode choisie n'a pas été la bonne, mais nous devons retenir son objet premier, qui reste la participation du plus grand nombre à cette élection. Certains de nos collègues ont d'ailleurs été réceptifs à cette proposition, mais l'ont finalement rejetée en raison de cette considération de forme ou pour des raisons politiques. Toujours est-il que nous devrons poursuivre nos réflexions parlementaires dans les prochaines années afin de moderniser les règles relatives aux opérations électorales dans l'objectif de garantir au scrutin toujours plus de participation, de sécurité et de sincérité. Le groupe RDPI votera les conclusions de la commission mixte paritaire.

La première est celle qui accompagne toujours une commission mixte paritaire lorsqu'elle est conclusive. Je ne m'y attarde pas, mais il est évidemment satisfaisant d'observer le Parlement travailler en bonne intelligence., ce projet ce projet ne devait d'ailleurs pas poser de difficulté majeure, puisqu'il procédait au toilettage électoral, tant nécessaire qu'habituel, qui précède l'élection présidentielle. Toutefois, lors de sa discussion en séance, nous avons eu la surprise de découvrir un amendement présenté par le Gouvernement qui donna lieu à de vifs échanges.

du scrutin. Sur le fond, nous avons souligné les inconvénients que représentait le dispositif dans l'état où il nous était présenté. Cela dit, nous demeurons ouverts au débat : c'est peut-être une idée à creuser ou du moins une piste de travail et de réflexion pour repenser l'organisation de nos scrutins et lutter contre l'abstention. Finalement, c'est du point de vue de la méthode que cet amendement nous a paru le plus surprenant. Comme pour toute compétition, qu'elle soit sportive ou politique, on ne modifie pas les règles du jeu la veille de la finale ! Vous le savez, j'ai déjà dit dans cet hémicycle mon goût pour le Top 14, ainsi que pour les valeurs que porte le rugby. Par conséquent, vous pourriez imaginer que je trouve beaucoup de défauts aux footballeurs ; il faut toutefois leur reconnaître au moins une qualité : ils savent parfois faire preuve de prudence et ne changent pas leur règlement avec légèreté. J'en veux pour exemple la méthode par laquelle ils ont institué l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR). Ce procédé fut d'abord autorisé à titre expérimental lors de matchs amicaux, été utilisé pour la première fois en compétition officielle en 2017 à l'occasion de la très peu disputée Coupe des confédérations. Qu'aurait-on dit si le premier test avait eu lieu, par exemple, lors de la Coupe du monde de 2018 ? Qu'aurait-on pensé d'une équipe de France championne du monde, mais victorieuse grâce aux aléas d'un test ? Dans des conditions équivalentes, que risquerait-on de dire d'un Président de la République élu au bénéfice d'une expérimentation contestable ? Comme pour tout, les premières fois sont rarement une réussite, et cette digression sportive me conduit à dire combien les lumières de l'expérience sont nécessaires. Il y a des sujets pour lesquels l'improvisation n'est pas de mise : l'élection à la plus haute fonction de notre République doit être planifiée et se dérouler sans accroc. Il y va de la confiance qu'accordent nos concitoyens aux institutions de la Nation. Ainsi, l'idée même de proposer et d'instituer ce vote anticipé par voie d'amendement, et pour la première fois à l'occasion de l'élection présidentielle, était de nature à nous interroger, voire à nous inquiéter.

Sur ces questions, il faudra peut-être évoluer dans les prochaines années, mais il ne paraissait pas opportun que cela ait lieu dès 2022. Dans ces conditions, le groupe du RDSE votera les conclusions de la

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi, qui aurait dû n'être qu'une routine législative précédant l'élection présidentielle, a pris une ampleur dépassant largement l'écho de ses faibles ambitions. Sans crier gare, sans débat ni étude d'impact, le Gouvernement a déposé un amendement visant à proposer le vote par anticipation la semaine avant l'élection présidentielle dans certaines communes dotées de machines à voter. à voter. Nous avons toutes et tous été pris de court par ce manque de sérieux du Gouvernement. Sur la forme, d'abord, puisqu'un tel dispositif impliquerait des moyens importants de sécurisation technique et juridique. Les risques de fraudes liés à l'usage du vote sur les machines ne peuvent être minimisés.

Nous nous félicitons donc que l'examen en CMP n'ait pas conduit à la réintroduction de cet amendement. Cet épisode nous aura cependant révélé une défaillance inquiétante dans les méthodes de travail de l'exécutif. À rebours de la logique du Gouvernement, nous estimons que la portée de la campagne électorale ne doit pas être minimisée. Nous souhaitons que l'ensemble des candidats puissent la mener dans de bonnes conditions et que les électeurs soient correctement informés. Cela nous paraît d'autant plus nécessaire en période de pandémie. C'est pourquoi nous avions déposé des amendements sur les sondages, par exemple, afin d'aller plus loin que la publication des marges d'erreur et de limiter la manipulation de l'opinion par un outil qui n'a rien de neutre.

Nous ne pouvons laisser la bonne information des citoyens entre les mains des grands groupes privés détenant les médias. Le rôle du législateur doit être de réguler l'organisation des échéances démocratiques afin de garantir des débats d'idées pluralistes et représentatifs de l'ensemble de la société. concernant la tenue de la campagne et de l'élection, face à la situation sanitaire dans laquelle nous sommes depuis maintenant un an, l'absence de dispositions pour anticiper les risques de perturbation nous paraît à contre-courant et dommageable. Nous sommes pourtant Le vote représente pour nous un pilier fondamental de la démocratie. Contre sa déterritorialisation et sa complexification par des artifices techniques, nous défendons la forme citoyenne du scrutin. Afin que chacune et chacun de nos concitoyens puisse participer pleinement à l'exercice du droit de vote, nous avions également déposé un amendement défendant la tenue de bureaux de vote dans les établissements pénitentiaires. Le texte de la CMP intègre des améliorations votées par le Sénat : sur l'accessibilité de la propagande pour les personnes handicapées, la publication des comptes de manière plus transparente ou encore l'avancement de la date de publication de la liste des candidats, que nous avions porté par amendement. Nous regrettons cependant que nos autres propositions n'aient pas été retenues. Ce projet de loi aurait pu permettre des avancées, mais il demeure un texte d'actualisation à la marge du cadre de l'élection présidentielle. Il passe surtout pour nous à côté de l'essentiel : la remise en question d'un régime hyperprésidentiel, avec un Parlement mis à distance. C'est pourquoi, vous le savez tous, nous nous inscrivons dans une démarche de révision de nos institutions pour aller vers une VI République véritablement démocratique et préservée des manoeuvres au service des ego et intérêts privés.

nous sommes réunis de nouveau pour examiner le projet de loi organique relatif à l'élection présidentielle, cette fois-ci à l'issue de son adoption en commission mixte paritaire. Je ne reviens pas sur la présentation technique du texte, dont le contenu est connu de tous dans cette assemblée. Lors de son examen au Sénat, le texte a été enrichi par plusieurs dispositions que j'estime, avec Philippe Bonnecarrère, dont je prends le relais sur ce texte, et le et le groupe Union Centriste tout à fait opportunes. Un point avait particulièrement retenu notre attention, c'est le dépôt d'un amendement gouvernemental visant à mettre en place pour l'élection présidentielle un vote anticipé au moyen de machines électroniques dans une liste limitée de communes dans chaque département. Le groupe centriste regrette que le débat ouvert par cet amendement sur un sujet aussi important n'ait pas pu être pleinement satisfaisant sur le fond. nous ne souhaitons pas écarter l'idée que ce sujet fasse à l'avenir l'objet d'une étude approfondie. Je pense qu'une réflexion, de manière sereine et transparente, autour des modalités opératoires des scrutins sera nécessaire dans les années à venir pour répondre

des élections locales en raison de la pandémie, il ne pourra pas en être de même pour une élection présidentielle. Au nom du groupe Union Centriste, je tiens à saluer le travail réalisé en commission mixte paritaire. nous félicitons que le texte, enrichi de nombreuses dispositions après son passage au Sénat, ait suscité l'adhésion sans réserve de la CMP. Notre est notamment satisfait du maintien des dispositions prévues à l'article 2 sur la durée de la période de financement de la campagne électorale, auxquelles il est très attaché. Le Sénat, en raccourcissant cette période à neuf mois au lieu de douze, souhaitait faire disparaître les incertitudes qu'aurait engendrées le chevauchement de deux périodes de financement de campagne électorale : d'un côté, les élections départementales et régionales et, de l'autre, l'élection présidentielle. Maintenant, les choses sont claires. Cette approche nous semblait nécessaire afin de prémunir les élus contre les difficultés de ventilation des dépenses entre ces différents scrutins. Ramener au 1 juillet 2021 le début de la période de financement pour l'élection présidentielle nous paraît être le moyen le plus simple et le plus efficace pour éviter tout débat et tout contentieux ultérieur. Par ailleurs, nous nous réjouissons du renforcement de l'accessibilité de la campagne électorale pour nos concitoyens en situation de handicap. Nous estimons qu'il s'agit d'une avancée pas seulement symbolique, mais véritablement majeure pour l'intégration et l'inclusion de tous dans la vie démocratique de notre pays. Nous partageons les mesures de bon sens s'inscrivant dans cette dynamique. À travers ce projet de loi organique, le Gouvernement poursuit la coutume qui prévoit, depuis 1988, que chaque élection présidentielle soit précédée d'une adaptation législative afin de conformer les règles de l'élection présidentielle aux évolutions de notre droit électoral. Ainsi, ce texte devrait avoir un impact limité, et c'est normal, dans la mesure où son ambition reste cantonnée à des mesures techniques qui ne bouleversent ni l'organisation de de l'élection présidentielle ni les règles de la campagne électorale. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe Union Centriste soutient le texte adopté par la CMP. La parole est à Mme

nous terminons nos travaux aujourd'hui par la discussion des conclusions de la commission mixte paritaire du 2 mars dernier sur le projet de loi portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République. Ce texte est essentiellement technique dans sa forme, comme l'ont reconnu les rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais il n'en est pas moins essentiel à la bonne tenue de la prochaine élection présidentielle, en 2022. en 2022. Ce scrutin occupe, depuis les premières années de la VRépublique, une place centrale dans notre ordonnancement institutionnel et politique. Les Français ne s'y trompent d'ailleurs pas, comme le montre le taux élevé de participation à chaque présidentielle. Le droit électoral applicable à cette élection est d'une telle importance qu'il est directement dérivé des articles 6 et 7 de la Constitution et prolongé dans une loi organique. Celle-ci nécessite cependant des mises à jour régulières pour demeurer en phase avec le droit électoral ordinaire. C'est ce qui a conduit à la quasi-systématisation du vote de lois organiques révisant le texte de 1962. Le présent projet de loi s'inscrit précisément dans cette démarche. Il a, par ailleurs, été heureusement travaillé dans un esprit d'échanges constructifs par nos deux assemblées. Concrètement, le texte dont nous discutons aujourd'hui comporte des dispositions fixant le délai imparti à la convocation des électeurs, complétant ainsi le texte jusqu'alors muet de la loi de 1962. Cela sécurise la préparation du scrutin. l'essentiel porte sur l'adaptation des règles pratiques applicables aux candidats et au scrutin. Il en est ainsi de la transmission des fameux parrainages, du vote des détenus, de la propagande électorale et, bien sûr, de la mise à jour des nombreux renvois du texte organique, demeuré statique, vers le code électoral, qui a évolué depuis la dernière présidentielle. À ce volet purement « hexagonal » s'ajoute un article consacré aux règles applicables aux Français de l'étranger, en particulier à leur vote par procuration et aux commissions de contrôle chargées de veiller à la régularité des listes électorales consulaires. Après sa transmission à notre assemblée, ce texte a encore pu être amélioré, en particulier grâce aux travaux de notre rapporteur. Le Sénat a, par exemple, adapté les règles de financement de la future campagne électorale, afin de permettre à celle-ci de se dérouler dans les meilleures conditions démocratiques et de transparence possible. C'est ainsi que les comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle seront disponibles en, comme c'est la règle pour les autres élections. Au-delà de ces mesures relevant plutôt de la technique pure, notre assemblée a aussi pris, sur l'initiative de notre collègue Philippe Mouiller, des mesures fortes en vue de garantir l'accessibilité de la propagande aux personnes à mobilité réduite. Le Sénat a enfin complété la mise à jour de plusieurs autres dispositifs concernant les parrainages ou encore les Français de l'étranger. À cet égard, je suis particulièrement satisfaite, en tant que sénatrice représentant les Français établis hors de France, de voir les 152 présidents des conseils consulaires rejoindre la liste des parrains. Dès l'automne 2018, j'avais demandé, avec mes collègues, que les conseils consulaires soient présidés par des élus pour respecter pleinement les principes démocratiques. Nous l'avons voté. Il était normal que les présidents de ces conseils puissent parrainer les candidatures à la présidence de la République. Avant de conclure, je ne peux négliger de mentionner le sujet qui a agité les débats dans cet hémicycle voilà trois semaines. Je fais référence à l'introduction tardive et maladroite par le Gouvernement d'une mesure portant sur le vote anticipé au moyen des machines à voter, introduction qui avait suscité notre vif étonnement. Je ne reviendrai pas ici sur les multiples fragilités constitutionnelles, juridiques et pratiques dont souffrait cette disposition, ni sur les interrogations soulevées par les méthodes de l'exécutif. Espérons Espérons au moins que cet intérêt soudain du Gouvernement pour les machines à voter l'incitera maintenant à prendre connaissance du rapport qui nous avait été confié sur ce sujet, avec mon collègue Yves Détraigne, en 2018. C'est à la quasi-unanimité que le Sénat a rejeté l'amendement du Gouvernement, et je me félicite de ne pas le voir figurer dans le texte dont nous discutons aujourd'hui. Dans ces conditions, le projet de loi organique, tel qu'il est issu des travaux de la CMP, nous semble satisfaisant. Le groupe Les Républicains le votera.

Le scrutin est ouvert.